La séance est ouverte bonjour chers collègues, bonjour monsieur le Ministre, le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué, il y a-t-il des observations, je n'en vois pas le procès-verbal est adoptée sous les réserves d'usage, l'ordre du jour appelle les réponses à des questions orales, la parole est donnée à ma collègue girondine Monique de Marco. Monsieur le Ministre, la dématérialisation des services publics s'accélère les confinements sont venues aggraver les fractures numériques si Internet facilite les démarches d'une majorité de Français, 13 millions d'entre eux rencontrent des difficultés, début 2021, dans le cadre du plan France relance le président, le précédent gouvernement a lancé des conseillers numériques, des contrats de projets de 18 à 24 mois, subventionné par l'État à hauteur du SMIG avec une formation, une certification, vous avez annoncé 4000 conseillers numérique auprès de 3000 collectivités locales et associations pour plus de 800000 accompagnement avec des ateliers collectifs ou individuels des déplacements au domicile des personnes les plus mobiles des conseillers numériques ont la capacité d'aller au plus proche des plus et des douaniers du numérique, le besoin continue d'exister, s'accroît. La formation n'a pas toujours été adopté au poste, le salaire est au minimum, leur situation est précaire aujourd'hui se pose la question de l'avenir de leur contrat, car ni les collectivités, ni les associations n'auront la capacité financière propres de les renouveler. Vous avez annoncé avoir mobilisé 75 millions d'euros pour la poursuite du dispositif dont nous n'avons pas trouvé la trace dans le PLF alors que 250 millions d'euros ont été nécessaires pour amorcer ce dispositif au vu de la baisse du budget annoncé comment l'État pourrait-il poursuivre à la même hauteur l'accompagnement financier des collectivités locales et des associations pour pérenniser ces emplois en 2023 et au-delà, je vous remercie. Merci, cher collègue, pour vous répondre, monsieur Jean-Noël Barrot Ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice le gouvernement par la voix de la première ministre, il s'est engagé dans une logique de pérennisation du dispositif des conseillers numériques France service l'État continuera donc d'assumer l'impulsion d'une politique de médiation numérique et financera ses missions sur plusieurs années après le temps de la relance, nous souhaitons que cette ambition soit véritablement collective qu'elle a ceci, tous ces acteurs et qu'elle les engage face à l'enjeu de société que constitue les fragilités numérique, nous devons construire une coalition nouvelle pour pérenniser l'action des conseillers numériques et plus largement celle de la médiation numérique s'agissant des conseillers numériques, je dois dire que je suis très optimiste après échange avec les parties prenantes à l'idée d'entamer cette phase qui suit la relance je sens tous les acteurs concernés par l'enjeu d'association de monter en charge du dispositif de meilleure organisation de l'action territorial des conseillers pour aller vers les publics fragiles, l'État va débloquer 44 millions d'euros de crédits nouveaux pour ce dispositif en 2023 qui viennent s'ajouter au crédit déjà provisionnés pour les contrats en cours, aboutissant sur une contribution de l'État de 75 millions d'euros et nous accompagnerons les coalitions d'acteurs locaux dans les collectivités dans la recherche de fonds complémentaires structurelles pour recruter et former plus de médiateur, les modalités de cette future politique seront concertés dans les prochaines semaines avec les parties prenantes, comme annoncé à Lens le 29 septembre afin de reconduire les contrats dans la durée, je souhaite par ailleurs vous rassurer sur un point : nous sommes en situation d'offrir une solution de reconduction des contrats qui arrivent à échéance d'ici le printemps dans les conditions actuelles, la formation a été un élément majeur du dispositif conseiller numérique, elle était obligatoire et certifiantes elle a permis de professionnaliser la filière mais a également mis en lumière une offre insuffisante, notre volonté est bien de faire monter en gamme, cet oeuf de formation, ce qui est aussi attendu sur le terrain, vous avez raison, nous en serons très prochainement avec le ministère du travail là une c'était la Mède num un engagement de développement de l'emploi et des compétences, concrètement, il s'agira d'un accord conclu entre l'État et les organisations partenaires qui vise à accompagner l'évolution des emplois et des qualifications. Merci, cher collègue, vous avez quelques secondes pour répliquer si vous le souhaitez. Donc, je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour ses informations et ses engagements. Merci, la parole est à présent à Madame Marie-Arlette Carlotti, pour poser sa question orale. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, ma question concerne la revalorisation des droits des élus d'arrondissement à Paris, Lyon et Marseille, si ces élus sont soumis aux mêmes règles aux mêmes obligations ont les mêmes responsabilités que tous les élus de toutes les communes de France, ils n'ont pas les mêmes droits pour l'essentiel les règles relatives aux conseillers d'arrondissements sont alignées sur celles qui s'applique aux conseillers municipaux, mais force est de constater que des inégalités perdurent dans l'acquisition de certains droits, notamment des droits relatives aux frais de garde au détachement au titre de mandat ou encore des droits relatifs à la forme inhumation et au bilan de compétences, aucun droit, non plus pour la prise en charge de dépenses d'accompagnement et d'aide technique pour les élus d'arrondissement qui sont en situation de handicap lors du débat sur la loi de finances rectificative de 2022, nous avons voulu souligner la nécessité d'introduire par la voie législative un alignement entre le régime applicable aux élus d'arrondissement et-ce et celui pour les conseillers de Paris et pour les conseillers de municipaux de Lyon et de Marseille, le groupe socialiste avait déposé un amendement à cet effet, et à cette occasion, ici même en séance, monsieur le Ministre, Bruno Lemaire, s'était engagé à reprendre cette proposition dans le cadre du projet de loi de finances pour l'année 2023, donc ma question Monsieur le Ministre, c'est est-ce que vous allez pouvoir tenir cet engagement et enfin vraiment enfin rétablir l'équité entre tous les élus locaux, merci. Merci, cher collègue, pour vous répondre, monsieur Jean-Noël Barrot Ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, vous me solliciter au sujet des droits des élus d'arrondissement et je vous en remercie tout d'abord, il doit être précisé que certains avantages des élus communaux, à l'instar des majorités des majorations indemnitaire et les majoration de la durée des crédits d'heures ne sont offertes qu'à certaines communes communes chefs-lieux communes sinistrées classée station de tourisme dont la population a augmenté suite à des travaux publics d'intérêt national comme une attributaires de la dotation de solidarité urbaine ou d'aménagement des communes d'outre-mer, si ces dispositions devaient être étendue au conseil d'arrondissement, elle ne leur serait donc pas systématiquement applicable de plus d'autres extensions davantage aux élus d'arrondissement soulève des difficultés opérationnelles à ce titre, l'ouverture pour le maire d'arrondissement et ses adjoints du droit à l'allocation différentielle de fin de mon doigt demanda la DSM se heurte au fait que cette allocation est financée par un fonds alimenté par les cotisations versées par les collectivités territoriales concernées, or les arrondissements ne sont pas des collectivités territoriales, distinctes de la commune et ne cotisent donc pas au fond de l'ADF. devrait être traités de la même manière car, en revanche ils sont élus, de la même manière vis-à-vis du suffrage universel de l'ensemble des citoyens, donc Monsieur le Ministre, regarder à nouveau si vous pouvez donner acte à ce que nous proposons, parce que c'est une vraie demande des élus locaux au moment où ils ont vraiment besoin d'être soutenus, merci. Merci, la parole est à présent à notre collègue le sénateur Monsieur Rémi Cardon proposé sa question orale. dévolue aux régions, soit un allégement fiscal de l'ordre de 7 2 milliards par an, le gouvernement a annoncé sa volonté de supprimer la part restante de CVAE destiné aux intercommunalités et aux communes, ce qui représente un nouveau manque à gagner de 7 milliards d'euros si cette suppression et et mise en oeuvre ce produit CVAE sera très probablement remplacé par un nouveau transfert de recettes de TVA aux collectivités territoriales, il s'agit là de la poursuite de votre processus d'érosion fiscale le de de fiscalité locale après la suppression de la taxe d'habitation et la réduction de la CVAE de de la CFE-pardon de collectivités sont victimes d'une recentralisation de leurs ressources, s'appuyant sur une philosophie néolibérale et qui ne croit pas à l'efficacité de la décentralisation comme si Monsieur le Ministre, les élus locaux n'étaient pas aptes à gérer leurs finances publiques la CVAE représentent environ 14 milliards, qu'il est d'ailleurs directement fléchée vers les collectivités locales et leur permet de faire fonctionner leur commune leur territoire mais également la l'exercice de leurs compétences, comme le social, l'activité économique, le transport ou encore l'éducation monsieur le Ministre de la question est la suivante : dans un contexte où le déficit public atteint des sommets, l'État est-il réellement capacité de supporter durablement une compensation intégrale et dynamique de la CVAE due aux départements et au bloc communal : comment garantir que la compensation ne deviendra pas rapidement obsolète et déconnecté de la réalité de l'activité de l'activité économique du territoire, je vous remercie. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur, Rémy Cardon, conformément aux engagements pris par le président de la République et le gouvernement, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sera totalement supprimée cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'objectif de soutien de l'activité économique et de reconquête industrielle elle poursuit l'allégement des impôts de production initiée en 2021, dans le cadre du plan de relance en cohérence avec la stratégie de maîtrise des finances publiques la CVAE sera réduite de moitié en 2023 et totalement supprimé en 2024 la perte de cette recettes induites par cette suppression sera compensée aux collectivités territoriales, dès le 1er janvier 2023 par l'affectation d'une fraction de TVA, le recours à une affectation de TVA permettra ainsi aux collectivités territoriales de bénéficier d'une recette pérenne et dynamique, qui évolue en lien avec l'inflation, notamment, par ailleurs, un amendement du gouvernement propose d'élargir la période de référence pour calculer la fraction de TVA affectée aux collectivités à 2023, il s'agit ainsi de tenir compte du dynamisme des recettes de CVAE que les collectivités auraient dû percevoir l'année prochaine, le montant de la compensation pour chaque collectivité locale sera ainsi déterminé sur la base d'une moyenne quadriennal de leurs recettes de CVAE année 2020, 2021 2000 22 et 2023 en outre l'incitation pour les communes et les intercommunalités à attirer de nouvelles activités économiques sur leur territoire, sera maintenu à cette fin, la dynamique actuelle de la fraction de TVA sera affectée à un fonds national d'attractivité économique des territoires dont les modalités de répartition, tenant compte du dynamisme économique de leurs territoires respectifs seront arrêtés à l'issue

les départements n'ont pas souhaité intégrer ce dispositif, par conséquent, chaque département bénéficiera de la dynamique de TVA associée à la fraction dont ils bénéficient sur le modèle de la fraction affectée aux régions depuis 2021, enfin, la perte de cette recette découlant de la suppression des frais de gestion de CVAE bénéficiant aux régions sera compensée à ces collectivités par l'institution d'une dotation budgétaire dont le montant sera égal au montant des frais perçus par elle en 2022. Merci monsieur le ministre, monsieur car, donc vous avez quelques secondes pour répliquer. écoutez Monsieur le Ministre, ce que je comprends, c'est la réalité, c'est que vous êtes en train de progressivement mettre sous tutelle les les collectivités tutelle financière, c'est déjà pas mal et puis, en plus de ça, c'est tout simplement les impôts des ménages qui vont financer les impôts de production, c'est bien ça le problème de philosophie Monsieur le Ministre. Merci, cher collègue, la parole est à présent un autre collègue sénateur Jean-Marc Todeschini proposé sa question orale. Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, la loi de finances rectificative pour 2022 prévoit des conditions cumulatives pour que les collectivités territoriales puissent bénéficier du dispositif de soutien, votée par les parlementaires, ainsi les collectivités doivent cumuler une épargne brute fin 2021 inférieur à 22 % de leur recettes réelles de fonctionnement et que c'était l'épargne brute connaissent une baisse de plus de 25 % sur l'année 2022, je voudrais aussi, je veux souligner que l'effet couperet de ces seuils cumulatif va laisser de très nombreuses collectivités en dehors de tous les dispositifs de soutien souhaitée par le Parlement, enfin les critères retenus peuvent permettre que des collectivités au potentiel fiscal élevé, voire très élevé mais à la gestion imprudente puisse se trouver aider quand des autres avec un potentiel fiscal très faible mais bien géré par leurs élus successifs ne recevront aucune aide ainsi l'indispensable augmentation du point d'indice ou plus encore le renchérissement du coût de l'énergie, comme des denrées alimentaires risque de du rêver très fortement les Budgets des secondes le potentiel fiscal par habitant supérieur ou non à la moyenne de la strate ainsi que l'effort fiscal ne serait-il pas des critères permettant une meilleure répartition des aides voulues par le Sénat aussi je vous demande quelles sont les solutions qui vous semble possible pour que ces collectivités au potentiel fiscal faible, particulièrement celles de taille modeste, ne souffre pas d'un traitement qu'elles ressentent comme inéquitable et puis son corps ne se retrouve pas dans des situations budgétaires très précaire au seuil de l'exercice 2023. Merci, cher collègue, pour vous répondre, monsieur Jean-Noël Barrot Ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Jean-Marc Todeschini, je vous remercie pour ces questions en ce qui concerne votre première interrogation au 31 décembre 2021 près de 24000 collectivités répondait au 1er critère d'éligibilité au dispositif institué par l'article 14 de la loi de finances rectificative du 16 août 2022, en ayant une épargne brute représentant moins de 22 % de leur recettes réelles de fonctionnement en ce qui concerne les seuils rendant éligible au dispositif, je me permet de préciser que l'article 14 de la LFR en impose 3 un seuil de fragilité financière représentée par le ratio entre l'épargne brute et les recettes réelles de fonctionnement en 2021 que je viens d'évoquer un seuil de situation financière dégradée pour les collectivités, subissant une perte d'épargne brute en 2023 supérieure à 22 enfin un seuil de capacité financière du territoire matérialisée par un potentiel financier inférieur au double de la moyenne de la strate démographique à laquelle la collectivité appartient ces seuils ont pour objet de concentrer le soutien de l'État sur les communes et les intercommunalités les plus fragilisés financièrement du fait de l'inflation, un soutien homothétiquement à toutes les collectivités n'est pas souhaitable car elle conduirait à un saupoudrage de la dotation et aurait pour conséquence un soutien moins important pour les collectivités établissements les plus affectées par l'inflation, enfin en ce qui concerne le critère de potentiel financier, il convient de souligner que ce dernier appréhende plus justement la richesse relative d'un territoire dans la mesure où le potentiel financier intègre, en plus du potentiel fiscal, le niveau de la dotation forfaitaire perçus au titre de la dotation globale de fonctionnement par ailleurs l'effort fiscal que vous évoquez, constitue aujourd'hui un indicateur financier contesté dans la mesure où la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales impose une redéfinition de ces paramètres, ainsi qu'en attestent les travaux du comité des finances locales menées depuis 2021, c'est pourquoi le gouvernement a retenu un critère d'éligibilité sur le potentiel financier pour cibler les collectivités territoriales, bénéficiaires du dispositif. Merci, monsieur le Ministre, chers collègues, vous avez quelques secondes. Merci madame la présidente, seul ministre, votre réponse ne peut être satisfaisante après après les annonces confirmée ce matin par le ministre du Budget, en faveur des entreprises qui, pour certaines souffrent énormément, réponse : non, ça dix faisant donc pour les collectivités, aujourd'hui elles dépendent en grande partie des dotations de l'État et pour les plus modestes, des communes, la dépendance est totale et mon collègue Rémi Cardon vient viens d'évoquer aussi la CVAE qui contribue aussi à une perte de de ressources. ressources. Propres des communes aujourd'hui, les maires ont la très nette impression que la libre administration des collectivités n'est plus vraiment une réalité vous allez tuer les collectivités qui représente près de 3 quarts de l'investissement public, si cela continue. Merci, cher collègue, la parole est à présent à notre collègue sénateur, monsieur Jean-Pierre Decool pour cette question orale. Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, le 10 mars 1964 la France, le royaume de Belgique ont signé une convention fiscale qui est toujours en vigueur aujourd'hui, cette convention pose dans son article 10 le principe que les revenus issus de la fonction publique sont imposables dans l'État payeur toutefois le paragraphe 3 de ce même article prévoit une disposition spécifique, si la personne concernée, travaillant dans la fonction publique possède la nationalité de son pays de résidence sans posséder la nationalité de l'autre État, en l'occurrence la Belgique alors sa rémunération sera imposable dans son pays de résidence en ce sens une personne travaillant en Belgique résidant en France et possédant la nationalité française, sans avoir la nationale il belge pourra voir sa rémunération issus de la fonction publique belge imposé en France ainsi cette disposition protège-t-elle les nationaux français d'une imposition belge 20 à 30 fois supérieurs afin d'éliminer la double imposition en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune pour prévenir de l'évasion et la fraude fiscale, une nouvelle convention a été signée le 9 novembre 2021, cette nouvelle convention retient sur cette disposition, en vigueur depuis près de 60 ans et prévoit désormais que les travailleurs français du secteur public doivent payer les impôts en Belgique les frontaliers français sont donc très inquiets de cette nouvelle réglementation, à un moment où la question du pouvoir d'achat ne peut être éludée, des centaines de familles sont concernées aussi, ma question est-elle simple : pouvez-vous apporter une réponse précise à cette situation, entendez-vous exclure de l'application de cette convention, le personnel public déjà embauchés avant la signature ou la ratification de la convention, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à présent au ministre Jean-Noël Barrot Ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Jean-Pierre de la France et la Belgique ont signé le 9 novembre 2021, une nouvelle convention fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, destiné à remplacer celle actuellement en vigueur, signé le 10 mars 1964 cette convention contient de nombreuses avancées, favorable à la France, elle préserve aussi le régime spécifique des frontaliers prévu au protocole additionnel à l'actuelle convention s'agissant des rémunérations de sources publiques la convention franco-belge signée le 9 novembre 2021 repose, sauf exception, sur le principe de l'imposition par l'État, qui verse ses revenus ce principe est logique car ses revenus publics sont financé par les ressources publiques publiques notamment fiscales de cet état, la rédaction de cette clause qui est conforme au modèle de l'OCDE se retrouve couramment dans notre réseau conventionnel et en particulier dans les conventions négociées récemment. Ceci explique que la nouvelle convention prévoit que les salaires des personnes travaillant en Belgique pour une entité publique belge soit taxé en Belgique, même si elle habitent en France l'inverse sera également vrai s'agissant des résidents de France, seule une catégorie de travailleurs verra son régime d'imposition modifié par les dispositions conventionnelles futur, il s'agit des résidents français possédant la seule nationalité française percevant des traitements publics de sources belges et exerçant leur activité en Belgique, ses revenus sont imposables en France en vertu des règles actuellement en vigueur et seront imposables en Belgique, par application de la nouvelle convention en 2021, comme vous le relevez il existe un différentiel entre l'impôt sur le revenu, belge et l'impôt sur le revenu français mais la législation en Belgique pourrait évoluer dans un sens plus favorable à l'avenir, le gouvernement belge a en effet proposé des pistes de réforme. Merci, monsieur le Ministre Monsieur de colle quelques secondes pour répliquer. C'est le dix, merci pour cette cette réponse à moitié satisfaisante puisque la décision appartiendra à nos amis belges, il faut tout de même que nous gardions l'esprit que, depuis 1964 les Français se sont sentis protégés par cette convention fiscale et on peut comprendre les craintes tout à fait légitime des familles transfrontalière, je vous remercie de donc de porter attention et avec bienveillance pour nos familles françaises. Merci, cher collègue, la parole est à présent hein, notre collègue, Madame la sénatrice Catherine Dumas. Merci madame la présidente, madame la ministre, j'aimerais attirer votre attention sur un projet qui a été initié par le président de la République de l'époque, en octobre 2016, un projet qui peine à se mettre en place, il s'agit du projet de la Cité du théâtre dans le 17ème arrondissement de Paris, ce projet est directement lié à la réhabilitation des Ateliers Berthier, cette cité du théâtre offrirait, Madame la Ministre, au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, au Théâtre national de l'Odéon et à la Comédie Française des capacités de représentation de stockage de répétition d'accueil du public, en cohérence avec leurs ambitions artistiques : internationale, nationale, voire municipal, un groupement d'intérêt public ayant vocation à conduire ce projet réunit d'ailleurs depuis 2019, ces 3 institutions culturelles ainsi que l'État, la ville de Paris à travers un voeu relatif à la reconversion des Ateliers Berthier en une cité du théâtre, adopté en conseil de Paris, à l'unanimité, fin 2021 a également montré son grand intérêt pour ce projet, le déménagement nécessaire des activités de l'Opéra Garnier était prévu et financé sur le budget 2022 la ligne budgétaire non utilisés, portée de 9 à 11 millions d'euros dans le budget 2023 alors Madame la Ministre est-ce le signe que ce projet de Cité du théâtre va enfin pouvoir se concrétiser pour la culture pour Paris et pour le 17ème arrondissement. Si la parole est à présent à madame Rima Abdul-Malak Ministre de la culture. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Catherine Dumas, alors oui, vous l'avez dit le projet de Cité du théâtre a été décidée en octobre 2016 pour porter au fond un nouveau projet pour ces 3 institutions réunis le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, le théâtre de l'Odéon, la Comédie-Française, un projet qui relie formation création diffusion dans un pôle commun ce projet a ensuite été confirmée par Françoise Nyssen, ministre de la culture en 2017 il a avancé, il y a une mission programmation un dialogue compétitif, qui a sélectionné la maîtrise d'oeuvre la création d'un GIP, un groupement d'intérêt public et la réalisation d'études par la maîtrise d'oeuvre mais mais mais voilà 6 ans après. Le coût n'est pas celui qui était fixé. En 2016 où on était à quatre-vingt-six millions hors coût du foncier, et voilà que aujourd'hui l'avant-projet sommaire qui a été remis par les architectes aboutit à 141 millions, soit un dépassement de 55 millions, hein, on a du coup missionner un expert indépendant pour qu'on puisse avoir peut-être des scénarios qui permettraient de revenir un peu plus proche de l'épure budgétaire initial, cet expert a proposé plusieurs pistes en réalité 4 scénarios qu'on a dû expertiser en lien avec les institutions concernées et nous prendrons une décision prochainement pour choisir un de ces scénarios en tenant compte de chaque avis de chacune des 3 institutions et de déchiffrage complémentaires qui ont été nécessaires, on aura aussi besoin de faire une évaluation précise des surfaces à acquérir auprès de la Ville de Paris, vous le savez, pour pouvoir aussi déterminer avec les services compétents la la valeur foncière associés pour le site Berthier, en tout cas merci de votre mobilisation, je sais que vous êtes nombreux à me parler régulièrement de ce projet emblématique qui nous tient à coeur, je pense aussi au maire du 17ème arrondissement Geoffroy Boulard la députée Caroline Yadan et bien sûr mon collègue Stanislas Guerini, avec qui j'en parlais encore hier donc. Nous nous sommes Madame la Ministre, pour chercher une solution, merci, vous avez quelques secondes. que vous avez bien voulu apporter en personne aujourd'hui, lors de cette séance de questions orales et je voudrais dire, hé bien, espérons que 2023 soit enfin la concrétisation de ce beau projet culturel pour Paris. Paris. La parole est à présent à notre code madame Chantal de scène proposé ça existe. Merci madame la présidente, madame la ministre ma question porte sur les difficultés que rencontrent les communes concernant les demandes d'autorisations d'urbanisme pour l'installation de panneaux photovoltaïques dans les zones classées bâtiment historique à titre d'exemple, la commune donnée sous Auneau l'est du département d'Eure-et-Loir, dispose d'un plan local d'urbanisme prévoyant les adaptations nécessaires pour tenir compte des objectifs de développement durable, prévue par les politiques publiques actuellement mises en oeuvre, or cette commune est classé bâtiment historique ainsi toutes les demandes d'autorisations d'urbanisme portant modification extérieure des bâtiments dans ce secteur sont soumises à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, les projets d'installation de panneaux photovoltaïques sur toitures ils font systématiquement l'objet d'un refus de l'architecte des Bâtiments de France lorsque l'Exposition est prévu plein sud, pourtant le choix de ce positionnement est liée à une meilleure Exposition au soleil permettant un rayonnement Direct et un rendement optimum ces avis se trouve ainsi en contradiction avec l'objectif, l'objectif affiché de développement des énergies renouvelables, pourtant la crise climatique et la crise énergétique rendent le développement des énergies renouvelables, nécessaire, madame la ministre, je souhaiterais savoir quelles mesures le gouvernement entend mettre en oeuvre pour encadrer les avis des architectes des Bâtiments de France afin qu'ils ne fassent pas obstacle au développement des énergies renouvelables dans les zones classées monuments historiques. Merci, cher collègue, pour vous répondre madame Rima Abdul-Malak Ministre de la culture. Madame la présidente, madame la sénatrice de Seine merci, vous mettez le doigt sur un sujet qui m'importe beaucoup, comment concilier la transition écologique, le développement des énergies renouvelables et la protection du Patrimoine c'est c'est très important et cette conciliation, au fond, elle est déjà au coeur des missions des ABF les Architectes des Bâtiments de France, puisque leurs avis ont pour objectif de préserver le Patrimoine et d'éviter au fond un caractère un peu disparates de certaines installations photovoltaïques, mais pas d'empêcher l'installation de panneaux photovoltaïques, en réalité, vous savez, les sites protégés, ça représente à peu près 6 pour 100 du territoire national et les refus des ABF sont absolument pas systématique, en réalité sur même très rare, si je vous prends les chiffres de 2021 les ABF, ils ont instruit pour l'ensemble du territoire français, plus de 515000 dossiers. 12800 dossiers. Porté sur des installations photovoltaïques, donc déjà que de 5 % parmi ces 12800 dossiers seulement 2300 ont fait l'objet d'un premier avis défavorable accompagné dans la majorité des cas de recommandations en termes d'emplacements de teintes je vous passe les détails techniques, mais certains ensuite ont pu aboutir, s'agissant donné sous sous dont vous parliez, la commune en Eure et Loir, j'ai vérifié de déclaration préalable, ont fait l'objet d'une instruction par l'ABF au titre des abords de monument historique en 2021 et 2022 pour l'installation de panneaux photovoltaïques et dans les 2 cas, l'ABF a donné son accord assorti de prescriptions, donc vraiment je pense que dans cette logique de dialogue, on peut arriver à trouver l'équilibre entre protection du Patrimoine et énergies renouvelables, on est en train de travailler actuellement sur une instruction ministérielle avec le ministère de la transition écologique pour donner un cadre aux ABF et aux collectivités pour s'y retrouver et voir quelles sont les bonnes solutions pour concilier les 2, merci beaucoup. Merci madame le Ministre, chers collègues, vous avez quelques secondes si vous souhaitez répliquer. merci madame la Ministre pour votre réponse, effectivement, il faut pouvoir concilier les intérêts patrimoniaux et les intérêts écologiques, il faut travailler à ce que il y ait des prescriptions qui permettent justement l'installation de ces équipements, parce que si on avait tenu les mêmes propos lors de l'électrification, par exemple, hé bien dans certaines endroits, nous n'aurions toujours pas l'électricité alors actuellement on a éventuellement des files qui cernent des des sites protégés remarquable avec le temps, on les enfouit je pense qu'on pourrait avoir des dispositions des préconisations similaire pour ce qui concerne les panneaux photovoltaïques. Merci, cher collègue, la parole est à présent hein Madame Hélène Conway Mouret. Merci madame la présidente, madame la Ministre notre réseau consulaire, pilier de notre service public, a perdu plus de 30 % de ses personnels en 20 ans, la création de 100 ETP en 2023 et donc une bonne nouvelle, il est notamment sorti fragilisé du programme Action publique 2022 en participant au tiers de la réduction de 332 emplois demander au ministère partout à l'étranger, j'entends le témoignage de ses agents, sur lesquels a été transféré une grande partie de la charge de travail des personnels non remplacés, il doit aujourd'hui rattraper les retards accumulés pendant les 2 années de pandémie, auxquels s'ajoutent les nouvelles demandes, malgré tous leurs efforts, donc, de nombreux pays, les prises de rendez-vous sont saturés, les délais d'attente peuvent atteindre plusieurs mois s'ajoute à cela des officines privées qui bloquent les créneaux ouverts pour les revendent ensuite, repoussant d'autant les rendez vous de celles et ceux qui se connectent au site officiel je suis régulièrement saisi par des compatriotes qui ne parviennent pas à joindre leur consulat, même en cas d'urgence, dans la majorité des pays où les postes sont supprimés, le standard téléphonique et où l'expérimentation du service France consulaire n'a pas débuté l'accueil téléphonique est reporté sur les agents dans tous les services, il semblerait que l'externalisation consistant à renvoyer les les appels des usagers de 13 pays vers un centre d'appels induit finalement de nouvelles dépenses en termes de personnel pour l'encadrement des salariés du prestataire assurée par le ministère, ainsi que la rémunération de celui-ci réalisons-nous vraiment les économies escomptées, nous avons un atout précieux : celui de posséder l'un des plus grands réseau diplomatique et consulaire du monde qui repose sur des professionnels de grande qualité, vendredi prochain s'ouvriront les états généraux de la diplomatie, ces créations de postes en 2023 sont-ils le signe d'une première étape d'un effort dans la durée et d'une transformation structurelle, je vous remercie. Madame la présidente, madame la sénatrice Conway Mouret je réponds au nom de ma collègue Catherine Colonna, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, confirme que les services consulaires ont fait face à une forte demande liée en partie à un effet de rattrapage, suite à la crise sanitaire pour faire face à cet afflux et améliorer le service rendu à nos concitoyens, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, poursuit ses efforts de modernisation avec notamment la poursuite de l'envoi postal sécurisé à domicile pour les passeports et la mise en place d'une nouvelle plateforme de rendez-vous 2023 verra également la mise en place d'un centre de soutien spécialisé qui va être basé à Paris et qui viendra en renfort ponctuel des postes dans lesquels un besoin aura été identifié le ministère veille aussi à ce que la modernisation nécessaires à l'amélioration du service aux usagers ne se fasse pas au détriment de l'accueil physique qui demeure bien sûr une priorité dans notre réseau attention, là je vais vous donner plein de chiffres, la dotation du programme 151 or titre de s'établit à 141,1 millions d'euros en crédits de paiement cette apparente baisse qui est de 0,9 millions d'euros en crédits de paiement par rapport à 2022 est principalement due à l'absence d'élections présidentielles et législatives en 2023 parce que c'est ça qui qui crée la la variation hors réélection le budget du programme progresse en fait de 12,6 millions d'euros avec, dans le détail, plus 10 2 pour l'aide à la scolarité plus un virgule, un pour le service France consulaire et plus un 1000000 d'euros pour les aides sociales

c'était bien là le le but de de ma question, aujourd'hui, nous avons des consulats en souffrance, nous avons des personnels en souffrance, je ne pense pas que l'envoi de task force que qui, enfin qui est prévu, soit la réponse, je crois qu'il ne faut pas oublier que nos consulats à la fois la porte d'entrée vers la France mais pardon également des services de proximité qui sont vendus et qui sont essentiels pour nos compatriotes. Merci, la parole est à présent notre collègue Madame Sylvie Robert proposé sa question. Merci madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, il y a un mois, nous étions nombreux à nous émouvoir qu'un quart de finale du tournoi de Roland Garros, opposant de légendes du tennis mondial ne soit pas diffusée en accès libre sur le service public comme c'est historiquement le cas mais en session de nuit sur une plateforme à accès restreint, dit : tu parles forme a finalement accepté de diffuser gratuitement le match au dernier moment d'ailleurs moyennant une récupération des données sur l'utilisateur, il n'en demeure pas moins que 20 % des Françaises et des Français n'ayant pas accès à un Internet résidentiel et ceux qui sont aussi victimes d'électronique, ça aurait été de fait exclu de cet événement, il s'agit malheureusement du dernier exemple d'un mouvement de fond plus global qui tend à privatiser les événements sportifs de grande ampleur, via un découpage, un système de découpage et de vente par lots, aux chaînes de télévision, lesquels sont de moins en moins en accès libre, si ce système peut permettre d'accroître les revenus issus de la diffusion des compétitions et rencontre bien sûr, il présente néanmoins un risque évident d'éviction des publics qui n'ont pas les moyens financiers ni technique d'accéder aux chaînes payantes, c'est ce qui si nous partageons toutes et tous la conviction que le Patrimoine sportif mondial français ne peut devenir l'apanage de celles et ceux pouvant simplement souscrire de multiples abonnements ni de celles et ceux ayant les ressources numériques suffisante en d'autres termes, un meilleur équilibre doit être trouvé entre viabilité d'un modèle économique dynamique, d'une part et accessibilité du plus grand nombre au sport, d'autre part, si le décret du 22 décembre 2004 en son article 3 défini une liste des événements sportifs d'importance majeure pouvant être diffusé sur un service de télévision en accès libre, sa liste pourrait être élargie plus substantiellement au regard de l'évolution en matière de droite retransmission des événements sportifs, seriez-vous favorable Madame la Ministre, à faire de l'accessibilité du plus grand nombre, un motif d'intervention en urgence de l'Arcom pour garantir la diffusion d'un événement sportif de grande ampleur sur une chaîne de télévision en accès libre, cette nouvelle prérogative cadreur et je pense parfaitement avec le rôle de régulateur qui est assignée à l'autorité, je vous remercie. Merci, cher collègue, pour vous répondre madame Rima Abdul-Malak Ministre de la culture. Madame la présidente, madame la sénatrice Sylvie Robert, j'en profite pour vous remercier pour votre engagement pour les bibliothèques également ma collègue Amélie Oudéa-Castéra m'a chargé de vous comme ce sujet concerne nos 2 ministères et le vrai sujet, vous l'avez posé, c'est cette fameuse liste parce que la protection des événements dits d'importance majeure est encadrée par le droit de l'Union européenne, il offre la possibilité de définir une liste d'événements qui bénéficie d'une protection particulière en vue de les rendre accessibles gratuitement, au plus grand nombre en France, c'est un décret de 2000 IV qui fixe cette liste, qui compte actuellement 21 Événement uniquement sportif, en fait, c'est la liste la plus longue en Europe en Union européenne plutôt voilà qui témoigne de l'importance, en tout cas que nous accordons à l'accès du sport pour tous, donc oui, le gouvernement est favorable à un élargissement et à une modernisation de cette liste pour y intégrer notamment les Jeux paralympiques et des événements sportifs féminin. Il faut pour cela passer par plusieurs étapes, le précédent gouvernement avait lancé une consultation publique sur ce sujet en début d'année et nous nous apprêtons à notifier cette liste modernisé, complété à la commission qui va devoir la valider, il est important de rappeler aussi que les droits audiovisuels représentent une part importante des ressources des acteurs du sport français, ils sont essentiels pour assurer la pérennité des événements et le développement du sport en France, à travers notamment la formation des jeunes, c'est tout l'objet de la taxe Buffet qui assure, comme vous le savez, une solidarité financière du sport professionnel vers le sport amateur, c'est pourquoi nous restons attentifs avec ma collègue Amélie Oudéa-Castéra au maintien d'un juste équilibre entre la disponibilité des offres à un coût raisonnable pour les téléspectateurs et le développement économique des ayants droit, voilà un équilibre à a toujours recherché cet équilibre ne s'est pas nécessairement dégradé d'ailleurs au cours des dernières années, si on regarde ce que dit l'Arcom dans son rapport du 25 juillet 2022, le poids des contenus sportifs diffusé en télé gratuite a en fait augmenté de 4,2 % il est passé à 5,4 % entre 2012 et 2019, soit une hausse de 1,2 % je vous remercie. Merci madame le Ministre, la parole est à présent à ma collègue girondine Madame Florence Lassaad. Merci madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, ma question porte sur la dégradation de la prise en charge des nouveau-nés placés qui, en raison d'un manque de personnel dans les pouponnières sont confiés à la protection de l'enfance et peuvent demeurer à l'hôpital plusieurs mois ces nourrissons souffrent d'une forme de dépression appelé qui apparaît dans le contexte d'un long séjour à l'hôpital ou d'un placement et qui peut être imputée à une carence affective ou à l'absence d'une figure d'attachement l'hospitaliser est un état dépressif avec régression physique et psychique qui se manifeste chez certains enfants séparés précocement de tout lien d'affection, ces enfants dépérissent progressivement tant physiquement que psychiquement ce trouble a été terrorisé dès 1946 par le psychanalyste René Spitz aujourd'hui en raison de l'augmentation des besoins, on assiste à un déficit de la prise en charge certains nourrissons avec des conséquences dramatiques dans le développement de ses enfants et dans leur future vie d'adulte, madame la Ministre, les professionnels de la petite enfance tire la sonnette d'alarme et explique cette situation par l'augmentation du nombre de mesures de placement, une crise de recrutement des professionnels, conjugué à une diminution du nombre de familles d'accueil qui par ailleurs vieillissant ne souhaite plus accueillir des enfants de moins de 3 ans, dans ce contexte de tensions, des places de tout petits enfants peuvent être laissés en protection de l'enfance est restée à l'hôpital plusieurs mois tandis que d'autres sont accueillis dans des pouponnières surchargés cette situation inhumaine est parfaitement inacceptable, qui plus est, pour des nourrissons qui sont déjà en souffrance Madame la Ministre, je souhaiterais savoir quels moyens humains et financiers, le gouvernement entend déployer en urgence pour améliorer la prise en charge et nouveau-nés placés. Merci, cher collègue, la parole est à madame Charlotte Caubel, secrétaire d'État chargé de l'enfance pour vous répondre. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les parlementaires, madame la sénatrice sénatrice Florence Lassaad, la prise en charge des enfants et notamment celle des plus fragiles, est au coeur de ma mission est une priorité pour le président de la République, le gouvernement et la majorité présidentielle avant toute chose, c'est vrai, le nombre d'enfants placés en France a augmenté ces dernières années de plus de 35000 enfants entre 2015 et 2020 et le département dans lequel vous êtes élu, la Gironde a connu une évolution tout à fait similaire, toutefois, il est difficile de répondre précisément à votre question sur l'évolution du nombre d'enfants à pouponnière, hélas, il n'existe pas de statistiques national sur ce sujet, ma réponse est évidemment totalement insatisfaisante, notamment pour travailler avec l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfance, autour d'un référentiel commun et d'un constat partagé je travaille actuellement sur ce sujet et des statistiques et de la prise en charge des enfants avec l'ensemble des pouvoirs publics pour que les pouvoirs publics disposent à l'avenir de chiffres rigoureux, le GIP en France protégée devrait nous permette d'ailleurs d'améliorer la situation, parce que je vous rappelle la protection de l'enfance, c'est une compétence décentralisée la situation complexe que vous évoquiez tout à fait importante n'est pas la même d'un département à l'autre, chaque département tant d'adapter en permanence son offre aux besoins du du territoire, c'est une compétence décentralisée, mais l'État est présent et doit continuer à l'être, notamment en accompagnant les territoires sur le volet de l'attractivité des métiers, le recrutement, la crise du recrutement dans tous les métiers du social, et particulièrement dans la protection de l'enfance est une de nos priorités, tant il impacte la qualité de la prise en charge de nos enfants, ce n'est pas uniquement une question de moyens, comme vous le savez nous avons étendu les revalorisations salariales du Ségur de la santé au au secteur de la protection de l'enfance, les familles, les assistants familiaux aussi été au 1er au 1er septembre mais c'est une crise de sens à laquelle nous devons répondre, nous avons sur les moyens financiers, apporter des réponses avec de la contractualisation, l'État sera aux côtés des départements et des professionnels pour continuer la protection de nos enfants et notre engagement à leurs côtés. Merci madame la Ministre, chers collègues, vous avez une poignée de secondes pour répliquer si vous le souhaitez. Merci madame la présidente, madame la ministre, ces enfants de viande devront des adultes placés et on voit terminer leur vie, certains dans des fois Didier d'accueil médicalisé, c'est ça le c'est ça leur destinée, c'est ça qu'il faut combattre absolument donner à ses enfants, qui ont déjà fragilisés par leurs conditions d'abandon ou de ou sociale, il faut vraiment leur donner une chance de vivre normalement et de devenir des adultes tout à fait apte à la vie commune. Merci, cher collègue, la parole est à présent un autre collègue sénateur, monsieur Patrick Chaize. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, ma question porte sur le plan d'évolution du site de Ionna, de l'Institut national des sciences appliquées, l'INSA de Lyon, vous savez au a et la plastique vallée sont historiquement un territoire d'industrie qui regroupe plusieurs filières d'excellence, aujourd'hui ce sont plus de 600 entreprises avec près de 10000 emplois qui constitue un pole Dance fort d'entreprises innovantes en plasturgie dès qu'elle émergent les noms des grandes entreprises de renommée internationale comme partout en France, les entreprises de la filière ont besoin de nouveaux talents, ceci pour répondre aux 3 enjeux auxquels la filière est confronté, celui de rester compétitif face à la concurrence étrangère, celui de former de nouvelles forces vives dans un marché de l'emploi particulièrement tendu et enfin celui de préparer les chefs d'entreprise de demain afin de relever ces défis, les acteurs se doivent d'ancrer les étudiants d'ingénieurs pour alimenter en compétences, les entreprises de la vallée, la présence de l'INSA sur le territoire une Nassia constitue ainsi un atout incontournable, avec qui les professionnels ont toujours travaillé, ce site est un élément stratégique de croissance partenariale dans le secteur industriel de la plasturgie, toutefois, force est de constater que l'INSA, la volonté de faire évoluer le cycle ingénieur de la plasturgie, avec d'une part, l'arrêt de la formation par alternance qui a été acté dès la rentrée de septembre 2021 et d'autre part, l'arrêt du cycle de formation actuelle en cours au profit d'une année optionnelle, il en résulte que le nombre d'étudiant INSA tend vers une domination une diminution par moitié dans ce contexte et alors même que le Campus du constitue un véritable outil haut de gamme au service de l'enseignement, je souhaite savoir, madame un Ministre si vous entendez agir pour que la formation ingénierie durable des polymères et composites ce rapidement mises en oeuvre, je vous remercie. Merci madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Patrick Chaize, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et Sylvie Retailleau son professeur profondément attachés à la prise en compte des spécificités du territoire et ont à coeur d'accompagner ces opérateurs dans une définition de l'offre de formation qui correspond qui correspond pleinement aux besoins des recrutements locaux, c'est la raison pour laquelle le projet de formation présentée par l'INSA Lyon a été élaboré à partir de l'analyse des besoins exprimés par les entreprises du territoire d'Oyonnax, notamment par l'intermédiaire de via le syndicat professionnel de la filière plasturgie et plasturgie et composite, il est important en effet que les étudiants domiciliés sur le site d'Oyonnax puissent bénéficier de formations plus diversifiée et répondant à leurs attentes, l'INSA Lyon qui est fortement engagé en faveur du développement durable et de la responsabilité sociétale qui irrigue tous les niveaux du cursus ingénieur permet à ces diplômés d'être en adéquation avec les besoins de la région, l'INSA Lyon envoie donc un message fort en faveur du développement de ce territoire, en adaptant son offre de formation et ses structures aux besoins des étudiants et des entreprises locales, nous pouvons nous en féliciter, sur la question précise, monsieur le sénateur, de savoir si le niveau diplôme peut être proposé en troisième année, au lieu de la 5ème année il appartient évidemment à l'institut de voir comment articuler au mieux cette offre, mais bien sûr, le ministère de l'enseignement supérieur et la recherche sera soucieux de l'accompagner au mieux afin de répondent toujours aux besoins du territoire merci beaucoup. 80 étudiants, on est passé à 35 et on craint que cela diminue encore si vous me le permettez, je vous proposerai de dire à votre collègue Madame Retailleau de venir sur place parce qu'on a vraiment tous les outils pour pouvoir faire en sorte de pouvoir donner une information de qualité sur site et je aux besoins des entreprises du site. Merci, la parole est à présent à notre collègue sénatrice Madame Monique Lubin proposé sa question orale. Merci madame la présidente, madame la Ministre, moi je vais vous parler aujourd'hui de ces 350000 personnes à peu près, qui ont travaillé entre les années 1985 et 1990 sur des contrats aidés, qu'on appelait les TUC, à l'époque, les travaux d'utilité collective aujourd'hui, ce sont des gens qui sont en train de préparer leur retraite et qui se rendent compte que étant donné qu'ils avaient à l'époque un statut de la fin de la formation professionnelle, des cotisations retraite n'ont pas été payés et donc aujourd'hui il leur manque un certain nombre de trimestres ou ou en tout cas la validation en espèces sonnantes et trébuchantes de ces moi avoir de ses années de travail, alors je sais que les services du ministère concerné ont été saisis à plusieurs reprises et que des réponses ont été apportées des réponses qui se réfère à un décret du 19 mars 2014 ou à la loi du 21 août 2003 mais en fait, le contenu de ces, de ces décrets ou de cette loi ne ne répond pas aux demandes et aux problèmes posés à ces personnes-là, donc, aujourd'hui, ma question est de savoir si on pourrait discuter de de cette question qui concerne, je le répète, 350000 personnes, ce n'est quand même pas énorme, mais ce sont des gens qui pour certains ont même rempli à l'époque, hein, des missions de service public auprès de certaines administrations, il faut le dire ou dans des communes et il me semble que se mettre autour d'une table et discuter d'une possibilité de valider financièrement ces ces, ces périodes-là, il me semble que ce serait une sacrée avancée merci madame la Ministre. Merci, cher collègue, pour vous répondre madame Charlotte Caubel, secrétaire d'État chargé de l'enfance. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Monique Lubin, oui les personnes recrutées entre 84 et 90 dans le cadre de travaux d'utilité collective, avait à l'époque, le statut de stagiaire de la formation professionnelle, conformément à un décret de 1984 dès lors la couverture sociale de ces stagiaires étaient assurés par l'État, il bénéficier d'une protection sociale contre tous les risques du régime légal selon les dispositions en vigueur les cotisations été calculé sur des assiettes et selon des taux de cotisation forfaitaire, ce qui ne leur permettait toutefois pas de valider, comme vous l'avez dit madame la sénatrice la totalité de ces périodes pour le calcul de la retraite, le nombre de trimestres d'assurance vieillesse validés au titre d'une année civile n'était pas établi en fonction de la durée de travail accompli mais à raison du montant de la rémunération annuelle soumises à cotisation le seuil de validation d'un trimestre était fixé à des cotisations équivalant à celle versée pour 200 heures de travail rémunéré au SMIC, seuil trop élevé pour valider l'ensemble des trimestres compte tenu des cotisations versées depuis le 1er janvier 2014, ce seuil a déjà été porté à cent cinquante heures du travail rémunéré au SMIC, toutefois, il convient de souligner que la loi de 2003 portant réforme des retraites a ouvert au titre des années incomplètes comme des années d'études supérieures, une faculté de versements de cotisations pour la retraite pour racheter des trimestres qui ont donc qui a donc été ouverte aux personnes Chuck concernés en tout et de quatre cause une nouvelle procédure visant à faciliter la validation de trimestres de manière rétroactive pour les anciens TUC nécessiterait une évolution législative, madame la sénatrice la concertation en cours menée par Olivier Dussopt qui m'a donné la parole aujourd'hui avec les partenaires sociaux sur le projet de réforme des retraites pourrait aborder concrètement cette question au sein du cycle dédié à l'équité et à la justice sociale. Que c'est bien de ça dont nous parlons, madame la sénatrice, merci, merci, chers collègues, il vous reste une poignée de secondes, merci à vous la parole est à présent à notre collègue la sénatrice Madame vivait Lopez. Merci madame la présidente, madame la ministre ma question ce matin a au manque criant de places, un institut médico-éducatif les IME et ses conséquences tant sur la vie des familles que sur le personnel enseignant, en effet, les parents confrontés à des situations de handicap de leur enfant peuvent après instruction d'un dossier administratif très lourd à monter auprès des services départementaux, voir leur enfant orienté un IME or très souvent aucune suite n'est donnée au dossier, faute de place, alors qu'il n'existe que 656 place dans le Gard, pas moins de 250 enfants sont concernés, aucune ouverture d'établissements ne semble pourtant envisagé cette situation est extrêmement difficile à vivre et lourde de conséquences pour les parents, mais également pour les enseignants, en effet, pour pallier ce manque de place, certains de ses enfants sont scolarisés en milieu scolaire et inclusif, parfois même en milieu ordinaire, ils bénéficient parfois aussi de dispositifs particuliers solution louable mais qui ne peuvent être envisagés comme des solutions satisfaisantes ni pérenne pour ses enfants qui ont des besoins spécifiques, force est de constater ainsi que si l'inclusion scolaire a fait des progrès ces dernières années des enfants en situation de handicap se trouve toujours dans l'attente s'inscrit scolaire, le gouvernement s'était pourtant engagé à la création de centres spécialisés pour ne laisser aucun enfant sur le bord du chemin incontestablement les efforts entrepris ne sont pas suffisants, quelle solution Madame la Ministre : envisagez-vous donc pour permettre à ses enfants la scolarisation et lesquels et les soins auxquels ils ont droit, je vous remercie. Merci, cher collègue, pour vous répondre Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées. Merci madame la présidente, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Ivette Lopez. le sens de l'histoire veut que nous fassions évoluer notre organisation pédagogique afin de mieux accompagner les élèves en situation de handicap, certains de nos voisins européens ont déjà tracé le chemin vers une scolarisation pleine et entière des enfants en situation d'handicap en milieu ordinaire et c'est la direction que nous souhaitons poursuivre bien sûr progressivement, nous réfléchissons et nous allons vers la meilleure manière de le mettre en place, en respectant tous les acteurs qui aujourd'hui accompagne ces jeunes, j'entends les critiques sur le manque de place pour de nombreux enfants qui sont encore sans solution et je mesure à quel point cela peut être difficile pour les familles, nous travaillons en lien étroit avec l'éducation nationale pour améliorer cette situation et proposer des solutions pour les élèves en situation de handicap, nous avons développé de nombreuses structures spécifiques pour accueillir ces enfants au sein de l'Éducation nationale, tels que les unités d'enseignement autisme en maternelle et en primaire, les dispositifs d'autorégulation les dispositifs institut thérapeutique, éducatif et pédagogique les d'ITEP multiplier le nombre d'Ulysse dans les établissements scolaires et bien d'autres dispositifs encore nous continuerons parallèle d'investir dans les établissements médico-sociaux en créant des places de façon régulière en 2023 environ 300 places sont créées pour les enfants en situation de handicap et surtout dans le même temps, plus de 1000 places seront créées pour les adultes qui pourront ainsi laisser leur place aux enfants dans ces établissements dédiés alors comme je vous le disais, le sens de l'histoire est à l'inclusion, nous devons donc poursuivre et renforcer le rapprochement de l'éducation nationale et du médico-social, nous avons déjà des exemples sur les territoires où l'inclusion est totale et où elle fonctionne et c'est dans cette direction, nous souhaitons aller avec la prochaine conférence nationale du handicap qui tracera l'acte de de l'école et de l'université inclusive merci. Merci madame la ministre, chers collègues, vous avez quelques secondes. Merci madame la ministre, pour votre réponse donc, je vais dire agissant agissons il est vraiment urgent et important : merci. Merci, la parole est à présent à notre collègue sénateur Monsieur Henri Cabanel. Si madame la présidente, madame la ministre, face à des parents, des parents employeurs peu scrupuleux qui ne payent par leurs salaires des assistantes maternelles se retrouvent en grande difficulté financière, alors que le tribunal leur a donné gain de cause en effet des employeurs perçoivent une allocation versée par la CAF, la prestation d'accueil jeune enfant qui ne peut être saisie en cas de procédure judiciaire entre par employeur est assistante maternelle, puisque l'article IV du code de la Sécurité sociale, précise que ces prestations familiales sont incessibles et insaisissable, sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de la locataire, les assistantes maternelles, pourtant, se retrouve sans solution, alors qu'il y a fraude, elles sont donc dans l'incapacité de récupérer leurs salaires dans un contexte de forte médiatisation de ce problème qui a révélé que des centaines d'assistantes maternelles ne sont dans ce cas, je souhaiterais savoir quelles mesures le gouvernement envisage de prendre pour garantir le salaire des assistantes maternelles et trouver une solution pour celles dont les salaires sont tu restées impayées. Chers collègues, pour vous répondre Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur Henri Cabanel, la question du versement d'un salaire dus par un employeur relève avant tout du droit du travail et ce sujet a été remonté plusieurs fois au ministère des solidarités ces dernières semaines, c'est pourquoi le ministère a contacté Lucena femmes pour dresser un état des lieux précis du sujet en l'état actuel de la réglementation, l'absence de dépenses effectives par un parent employeur n'ouvre pas droit au versement de la prestation, dans le dispositif Pajemploi sans versement effectif du salaire est constitutif d'une fraude et donne lieu à la récupération des sommes indûment versées, il s'agit d'un garde-fou indispensable contre les impayés l'Urssaf a mis en place égale le monde depuis mai 2019 un service optionnel et gratuit appelé page emploie plus ce service assure le versement de la rémunération sur le compte bancaire du salarié dans un délai de quatre jours suivant la déclaration sociale de la famille Pajemploi prélève parallèlement sur le compte bancaire des parents employeurs la somme restant à leur charge, ce qui permet de simplifier et sécuriser les démarches toutefois la confiance, ce n'est pas tout à fait acquise entre par j'emploie plus et les assistantes maternelles, dont les représentants ne réclame pas une ni moment sa systématisation ceux-ci observe par ailleurs que la présence d'un intermédiaire ne change rien en cas d'insolvabilité les représentants d'assistants maternels ont fait remonter la situation de professionnels, privé de rhume, revenu d'activité et il y a le monde du fait d'une suspension d'agrément à titre conservatoire, ils insisté sur les conséquences lourdes pour le professionnel et sa famille, et ce alors même que l'instruction peut conclure à l'absence d'un comportement inapproprié, c'est pour ces raisons que le comité de filière, petite enfance constitué début 2022 a prévu de travailler sur la constitution d'un éventuel fonds de garantie des salaires dédié aux professionnels de l'accueil individuel cette piste de travail et celle qui étaient portés d'ailleurs par le syndicat Unsa-pro ce et je crois que, voilà, nous vous le voyez, ce sujet fait l'objet d'un suivi attentif du gouvernement et en particulier de Jean-Christophe Combe. Si Madame la Ministre, chers collègues, vous avez près d'une minute pour répliquer. Merci madame madame madame la Ministre de cette réponse, mais vous avez évoqué effectivement les prévisions pour empêcher ce qu'il arrive aujourd'hui des salaires impayés, moi j'aimerais que revenir sur les assistantes maternelles aujourd'hui qui sont dépourvus, parce qu'elles n'ont pas été payé par ses employeurs peu scrupuleux et ses employeurs presque plus le on fait une fraude à la CAF puisque ils ont touché quand même donc l'aide versée par la CAF, donc il faudrait vraiment que l'on puisse trouver une solution pour puisse pour que pour que la la CAF puisse récupérer ses fonds et au moins versé ces fonds aux assistantes de maternelles qui n'ont pas de salaire, aujourd'hui effectivement la leçon engagée devant les prud'hommes, donc des poursuites, elles ont gagné, mais elles se trouvent complètement dépourvu parce qu'elle serait obligée d'engager des frais supplémentaires d'huissier pour pouvoir récupérer les sommes qui apparemment donc risque de ne pas être récupérée, donc il faudrait absolument que le gouvernement Vienne à leurs côtés pour essayer donc de retrouver un minimum de salaire qui ont été payés. Merci, cher collègue, la parole est à présent à notre collègue sénatrice Madame Catherine Procaccia. Merci madame la présidente bonjour madame la ministre ma question porte sur les concentrations de dioxine qui ont été enregistrés auprès de l'incinérateur d'Ivry du sitcom en début d'année, c'est une étude menée par un collectif écologique qui avait révélé des concentrations anormalement élevé de dioxine tout autour de cet incinérateur qui est le plus grand d'Europe et qui brûle près de 730000 tonnes d'ordures par an, en février, l'ARS a recommandé aux habitants des communes proches, c'est-à-dire de Paris mais aussi du Val-de-Marne, de ne pas manger d'oeuf de poules élevées en plein air, la consommation régulière 9 pollué aux dioxines présentant des forts risques pour la santé, elle a aussi demandé une analyse toxicologique des experts cependant l'usine du comme dit toujours respecter strictement les normes en matière de rejets et elle est soumise à de nombreux contrôles lorsque j'ai posé ma question, madame la ministre au début de l'année, au ministre de la Santé, je souhaitais savoir dans quel délai, les résultats seraient connus et comment pouvait être évalué le lien entre l'incinérateur et les dioxines, je je n'ai pas eu de réponse, d'où la fais ce que je la pose maintenant 6 mois après, à l'oral, et j'aurai insiste sur la deuxième partie de ma question si l'usine n'est pas à l'origine des dioxines, quelles mesures concrètes, les instances environnementales et sanitaires compte prendre pour protéger la population parisienne et 22 marnaise. Merci, cher collègue pour vous reprendre Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées. Merci madame la présidente, madame la sénatrice Catherine Procaccia. Je vous prie d'excuser le ministre de la Santé qui m'a demandé de vous répondre aujourd'hui, mais il ne pouvait être là, néanmoins j'ai j'espère avoir les bonnes réponses, la surveillance des des émissions des incinérateurs, relève de la compétence de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'Aménagement et des Transports là de rillettes, les dioxines sont un paramètre systématiquement et régulièrement contrôlées les questions d'Exposition environnementales mises en lumière dans les analyses d'oeuf autour de l'incinérateur d'Ivry dans l'étude de la Fondation iWatch Watch, font l'objet d'un travail commun de la DGS et de l'ARS Île-de-France avec les agences sanitaires nationales cette étude avait révélé des niveaux de contamination des oeufs, dépassant les seuils réglementaires de commercialisation, l'ARS, dès qu'elle a eu connaissance de ces résultats a émis une recommandation de non consommation des oeufs d'élevage domestique dans la zone de l'étude, cette recommandation a été prise à titre conservatoire et prudentielles dans l'attente d'une évaluation plus approfondie, en effet, aucun lien de causalité n'a pu être établi par Tocci iWatch entre l'incinérateur et les résultats des prélèvements, ce point est confirmée par l'eau ensuite un groupe d'experts de la DGS a constaté que l'étude Tocci Watch souffre de défauts méthodologiques dont un manque de clarté sur les protocoles de prélèvement et d'échantillonnage et de plus, les études de lancer et de santé publique France souligne que résider à proximité de zones industrielles et d'incinérateurs ne semble pas modifier les niveaux d'imprégnation en dioxines à l'exception des populations qui consomment des produits issus d'animaux élevés dans une zone connue comme polluées, donc l'ARS lance une étude supplémentaire pour vérifier l'alerte de Tox Watch et déterminer s'il convient de maintenir la recommandation de non consommation des rencontres régulières ont été organisées avec différents acteurs dont le collectif trois heures et les résultats de l'étude sont attendus au 1er semestre 2023. Merci madame la ministre, chers collègues, vous avez quelques secondes pour répliquer. Merci, si je comprends bien, madame la ministre, il est recommandé de ne pas manger de boeuf élevé chez particulier en en milieu dense urbain, il ne doit pas en avoir énormément, mais ce que je regrette, c'est qu'on a déjà eu des premiers résultats au mois de juillet, qu'on les a pas communiqué qui a une population qui est inquiète inquiète cette inquiétude, on aurait pu la faire tomber et surtout ce que vous venez de le dire sur l'évaluation de l'analyse faite par un collectif peut-être dire tout haut que les la méthodologie n'était pas forcément la bonne. Merci, cher collègue, la parole est à présent à notre collègue sénatrice Madame Françoise Férat. Merci madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, ma question concerne l'extension du nutriscore aux fruits et légumes frais, comme vous le savez le Nutri score est un système d'étiquetage nutritionnel créée par Santé publique France afin de faciliter l'information et orienté le choix des consommateurs vers des aliments de meilleure qualité nutritionnelle, les bénéfices pour la santé, de la consommation régulière de fruits et légumes sont largement démontré consommer quotidiennement des fruits et légumes, joue un rôle positif dans la prévention des maladies telles que l'infarctus l'hypertension artérielle ou de nombreux cancers par la consommation des fruits et légumes reste encore très insuffisante sur les enfants et les adultes, nous sommes loin des 5 fruits et légumes, conseiller chaque jour le Nutri score étant un étiquetage reconnu et apprécié des Français, je demande simplement au gouvernement son extension aux fruits et légumes frais ah, hormis la noix de coco, qui est en classe B, ils le sont tous, je vous remercie. Merci, la parole est à présent à Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées pour vous répondre. Merci madame la présidente, madame la sénatrice Françoise Ferrat. Le Nutri score fait l'objet d'un soutien fort des consommateurs qui sont près de 94 % a déclaré être favorable à sa présence sur les emballages, les industriels décide de la poser sur leurs produits afin d'accroître aussi l'information et la transparence auprès des consommateurs, début 2022, ils étaient déjà plus de 875 à être engagée dans la démarche alors afin de renforcer cette information nutrition nutritionnelles au consommateur et d'encourager le choix d'aliments plus sains, le 4ème programme national nutrition santé prévoit d'étendre sur la base du volontariat, le Nutri à la restauration hors foyer, d'une part et aux denrées non préemballés d'autre part, le gouvernement travaille actuellement à l'élaboration d'un cadre juridique et opérationnel qui permettra d'étendre lu ça l'usage de ce logo Nutriscore sur la base volontaire aux aliments non-préemballés dont les fruits et légumes frais ainsi une consultation des parties prenantes, regroupant les représentants des industriels et des distributeurs, les administrations et santé publique France est menée depuis un an afin d'élaborer les conditions d'application du nutriscore sur ces aliments l'objectif bien sûr, c'est que le consommateur puisse disposer d'une information nutritionnelle simples, claires et transparentes dans les rayons de produits bruts, tels que les fruits et légumes ou les silos de vrac ainsi l'affichage du Nutri score en très grande majorité à pour les fruits et légumes permettra d'encourager la consommation de ces produits frais de bonne qualité nutritionnelle essentiels à un bon à un bon état de santé et, bien sûr, il faut poursuivre, encore et toujours les recommandations générales nutritionnelle, publié par la santé publique France qui encourage la consommation d'au moins 5 fruits et légumes par jour, je vous remercie. Merci madame la ministre, chers collègues, vous avez une petite minute. Pour oui merci madame la présidente, merci, Madame la Ministre, pour cette réponse qui qui est de nature à nous rassurer effectivement je, je le rappelle, c'est un un projet qui ne coûtera rien aux finances publiques, ni aux entreprises, et qui a un impact positif sur la santé, vous venez de de le rappeler, vous-même et il est immédiatement repéré par les consommateurs, vous êtes sans doute nombreux ici à avoir repéré sur des sur des sachets sur des paquets, une multitude de logo, le fait que ce nutriscore soit poser c'est vraiment celui qui est le plus facilement repérés, il est particulièrement incitatif et il sera de nature à favoriser la la filière des légumes et des fruits merci beaucoup. Merci, cher collègue, la parole est à présent à notre collègue sénatrice Madame à talons. Merci madame la présidente, madame la Ministre, en France, le diabète provoque 30000 décès chaque année, l'épidémie accélère et se sont actuellement 3 5 millions de diabétiques qui sont quotidiennement traitées par médicaments, soit 5,3 % de la population et aujourd'hui même, comme hier ou demain, 400 nouveaux cas auront été déclarés, mais surtout on estime qu'entre 500 et 800000 personnes sont porteuses de la maladie et l'ignore, face à l'ampleur de cette épidémie touchant plus particulièrement les jeunes, les campagnes de dépistage et de prévention sont indispensables, de plus, le moment du dépistage et l'occasion de partager avec le public, les connaissances sur le diabète et de développer la prévention de proximité des associations comme Agir, qu'on me contre le diabète qui intervient en Ardèche méridionale mène ses opérations avec des équipes composées de professionnels de santé et de bénévoles or seuls des professionnels de santé, tels que les médecins, les infirmiers, les armes, les pharmaciens et les sages-femmes peuvent légalement réalisé les dextro, ces prélèvements capillaires effectués lors des campagnes de dépistage, hélas, le manque de disponibilité des infirmiers bénévoles conduit ces associations à devoir limiter leurs actions, avec pour conséquence des retards dramatiques dans la prise en charge des nouveaux malades. Cependant, si les agences régionales de santé pouvait délivrer des dérogations, certaines associations pourrait pallier le manque d'infirmiers en continuant à pratiquer des dextro, des bénévoles du Mans, formé par des médecins diabétologue pourrait ainsi dépister massivement en autonomie, madame la ministre, je vous demande donc si vous envisagez d'aménager le droit en vigueur ou d'autoriser par voie réglementaire les ARS à déroger afin de ne pas retarder le dépistage de nombreux diabétiques, je vous remercie. Merci, cher collègue Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées va vous répondre. Merci madame la présidente, madame la sénatrice Anne Van allô. En France, la prévalence du diabète traité par un médicament était estimé à 5,3 pour 100 de la population en 2020, soit plus de 3 millions et demi de personnes la fréquence du diabète continue aujourd'hui de progresser, c'est un enjeu majeur de santé publique, vous l'avez dit, la fréquence du diabète de type II a augmenté de 0 9 % par an chez les hommes et de 0 4 % par an chez les femmes de plus de 45 ans entre 2010 et 2017, tandis que l'incidence avait diminué sur une période 2012, 2017 moins 2 virgule six chez les hommes et 3 9 moins de 3 9 chez les femmes, alors le diabète de type 2 évolue souvent en silence, car la glycémie augmente très progressivement un dépistage ciblé est recommandé tous les 3 ans chez les plus de 45 ans ayant au moins un autre marqueur de risque du diabète excès pondéral hypertension artérielle cholestérol antécédent familial, la mesure de la glycémie peut s'effectuer dans un laboratoire de biologie médicale par prise de sang chez soi avec des appareils de diagnostic rapide la mesure au laboratoire étant plus fiable et précise le maillage territorial en laboratoire permet quand même aujourd'hui un accès simple ainsi les pharmaciens d'officine sont autorisés depuis 2016 a réalisé dans le cadre des campagnes de prévention des tests capillaires d'évaluation de la glycémie, les possibilités d'accès au dépistage sont aujourd'hui nombreuses et le gouvernement n'entendent pas mobiliser de nouveaux acteurs, mais en même temps, rares renforcer sa stratégie de prévention du diabète, notamment au travers des rendez-vous prévention pris en charge à 100 % aux âges clés de la vie dès 2023. Merci madame la Ministre, la parole est à présent notre collègue Madame Sabine 20. depuis la fermeture de l'usine en 2003, il n'y a pas eu de campagne de détection du saturnisme infantile menées de manière systématique de nouveau alerté par les associations et les élus, l'État s'est enfin décidée en juin, a engagé une campagne de détection des cas de plombémie autour de Metaleurop, la campagne devait concerner 7511 enfants sur le périmètre du pic à Courcelles Les Lens : ma maison pardon Dourges le euphorie Noyelles-Godault, mais seuls 1200 enfants ont été testés, soit 12 % de la population cible, 8 enfants sont atteints de saturnisme et 68 doivent être surveillés, c'est extrêmement inquiétant, 8 enfants, la répartition des cas de saturnisme démontre que la pollution des sols contaminent les enfants depuis les jardins et les pelouses des maisons particulières dans les zones un et 2 du Pigs sur 200 hectares autour de l'ancienne usine polluée, entre 500 PPM et plus de 1000 PPM de plomb mais cette pollution des sols semble aussi contaminés : les enfants depuis une troisième zone de 400 hectares autour des 2 premières du Pigs cette zone identifiés par l'Ademe, dès 2011 comme pollué et pourtant soumise à aucune information particulière, il n'y a aucune servitude constructives de la part de l'État, les constructions, ils sont ainsi libres dans une zone polluée qui expose la santé des enfants, Madame la Ministre, quand l'état va-t-il enfin prendre la mesure de ce préjudice écologique et supprimer les sources de pollution issue de l'usine, Metaleurop en prenant à sa charge, comme c'est demandé depuis longtemps le décaissement et le remplacement des sols pollués merci. Merci Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées va vous répondre. si l'arrêt de la. Activité industrielle en 2003 a mis fin à l'émission de particules contaminées sur le site Metaleurop, les 5 communes limitrophes sont concernés par une pollution au plomb et vous l'avez dit, dès la fin des années 1990 de nombreuses actions de dépistage et d'information ont été menées le dépistage individuel sur ce territoire est en permanence accessible, en plus des campagnes collectives et en mai dernier, le préfet du Pas Pas-de-Calais a reçu les élus municipaux concernés pour lancer une nouvelle campagne de dépistage et les proposer depuis le 15 juin aux enfants et aux moins de 18 ans, cette campagne qui a fait l'objet d'une large information se poursuivra jusqu'au 7 novembre et prise en charge à 100 % bien sûr pour les moins de 18 ans et les femmes enceintes au 10 octobre c'était 1000 100 40 enfants qui ont déjà participé soit, soit un taux de participation de 15 % que je peux trouver moi aussi trop faible 8 enfants présentant une plombémie correspondant au seuil de définition du saturnisme, soit 0,7 pour 169 enfants ont des résultats correspondant à un seuil de vigilance chaque dépistage positif fait l'objet d'une déclaration obligatoire qui déclenche une investigation environnementale pour traiter les sources et limiter l'Exposition, les familles des 8 enfants positifs ont été contactés par l'ARS et ont fait l'objet d'une visite au domicile pour mener ses investigations, une information sur les sources d'Exposition et les règles d'hygiène est en cours pour les familles des 69 enfants concernés par le seuil de vigilance, mais le gouvernement et et je crois qu'il faut que nous soyons tous derrière cela incite les populations au dépistage et c'est en fonction voilà de de ce dépistage que nous pourrons être encore plus efficaces pour, hé bien, la prévention et agir pour les accompagner. Collègues il faut une poignée de secondes. Oui, Madame la Ministre, vous n'avez pas complètement répondu à ma question, en tout état de cause, ça n'a, ça n'a que trop duré, c'est à l'État qui a laissé à l'époque et en connaissance de cause, cette usine polluée de réparer ce préjudice écologique et sanitaire, La parole est à présent à notre collègue sénateur, monsieur Olivier rythme. Merci madame la présidente, madame la Ministre, comme vous le savez, la répartition des chirurgiens dentistes sur l'ensemble du territoire est inégal et elle ne permet donc pas de garantir une offre de soins homogène, le département de la Haute-Saône subit tout particulièrement cette mauvaise répartition géographique, comme le souligne d'ailleurs les conclusions présentées par l'Observatoire national de la démographie des professions de santé, en novembre 2021, la densité moyenne européenne est de 74 dentistes, chirurgiens dentistes pour 100000 habitants, la densité nationale française et de 63 chirurgiens dentiste pour 100000 habitants, or 12 départements français ont une densité en chirurgiens dentistes inférieur à quarante dont la Haute-Saône. Dans certaines zones de ce département, dans le Nord, Haute-Saône, les bassins luxe oh vient lurons et Ju C1 l'écart de densité se creuse encore davantage pour atteindre moins de la moitié de la densité nationale. Pour paraphraser le président de la République lors de son intervention au congrès de la Mutualité, en septembre dernier, je cite, cette situation n'est pas acceptable, et elle le sera d'autant moins que la demande de soins augmente avec le vieillissement de la population, l'amélioration du système de la prise en charge financière mais aussi et surtout, réjouissons-nous en l'essor de la prévention de la santé bucco-dentaire. Dans le contexte très préoccupant que je viens de décrire l'actualisation du zonage des chirurgiens dentistes reporté à de multiples reprises s'impose dans les plus brefs délais pour rétablir l'accès aux soins, j'en viens donc à ma question, madame la Ministre quand cette actualisation du zonage sera-t-elle annoncé et surtout dans l'attente autori vous autorisez-vous l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté, en concertation avec l'ensemble des parties prenantes d'actualiser la carte des zones d'accompagnement régionale, je vous remercie. Merci, cher collègue, j'invite Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées à vous répondre. Merci madame la sénatrice Monsieur le Sénateur, rillettes, Matt le. Vous appelez vous appelez notre attention sur le zonage des chirurgiens dentistes en Haute-Saône, dans un contexte de tensions sur l'offre en soins dentaires qui malheureusement est aussi nationale mais plus importante dans votre, dans votre région, comme vous le signalez, dans l'attente des prochaines négociations conventionnelles et afin de favoriser l'installation des chirurgiens dentistes, là où les besoins sont les plus importants avant l'exemple de l'ARS Bretagne qui a fait le choix de compléter la cartographie actuellement opposable du zonage des chirurgiens dentistes par un ciblage de nouveaux territoires identifiés comme déficitaires, les zones d'accompagnement régionales en Bourgogne Franche-Comté, un autre choix a été fait, celui de ne pas proposer l'ajout de zones complémentaires afin de ne pas brouiller les informations données aux professionnels dans l'hypothèse où les zones identifiées par l'ARS s'avérerait et ne pas être les mêmes que celles qui sont identifiés dans le cadre de la révision nationale à ce jour, le jaune, le zonage médecin sert de référence, conformément à la doctrine nationale pour les contrats d'engagement de service public, chirurgien dentiste ce zonage de 2014 s'applique pour les aides conventionnelles de l'assurance maladie, alors dans l'attente de cette révision nationale l'ARS Bourgogne-Franche-Comté consciente des difficultés à tout de même ouvert la porte à certaines souplesses elle accepte d'accompagner après analyse des situations, les nouvelles installations et prend en charge les demandes d'aide exceptionnelle sur le fonds d'intervention régional pour favoriser l'implantation ou l'équipement dans une zone qui qui n'est actuellement pas classé comme sous-dense dès lors qu'un besoin s'avère justifiée. Merci, la parole est à présent à notre collègue sénateur monsieur Bruno Belin merci madame la présidente. Madame la Ministre, on le voit encore ce matin par les questions de nombreux collègues, le sujet des déserts médicaux interroges tous les élus et et je sais que vous même être mobilisés en Nouvelle, Aquitaine ou dans votre département des Landes, voilà c'est tous les sujets sur tous ses territoires nous reviennent tous les jours, alors le Sénat la semaine dernière a adopté une proposition de loi à l'initiative du président Retailleau, très bien, on essaye d'avancer, on sait très bien que cette proposition de loi donnera des effets que dans quelques années. Et pourtant, il existe aujourd'hui des outils législatifs, je pense à la loi du 24 juillet 2019 dont on attend toujours le décret d'application, alors quand on est dans une telle pénurie et on se demande bien pourquoi des décrets d'application ont du mal à venir, on nous avait ça avait été l'objet d'une question d'actualité au gouvernement en avril début de de l'année, on nous avait promis une arrivée de ce décret pour avril ça correspondait évidemment un calendrier électoral qu'on a tous en tête, donc ma question est simple Madame la Ministre quand le décret d'application qui permettra les stages d'internes en milieu rural, sera-t-il signé conformément à la loi du 24 juillet 2019. Merci, chers collègues, je vous invite, madame Darrieussecq à répondre à ce sénateur de votre région. Merci madame la la présidente, monsieur le sénateur Bruno Belin. Bon, la mesure sur laquelle vous m'interrogez et d'application immédiate. La maquette de formation du diplôme d'études spécialisées de médecine générale a été adaptée, elle prévoit que les étudiants en face d'approfondissement, accomplissant ce stage en soins en soins primaires autonomie supervisée auprès de maître de stage agréé à titre principal en en médecine générale, ils peuvent accomplir ce stage cette d'application immédiate, la loi du 24 juillet 2019 relatives à l'organisation à la transformation du système de santé prévoit en effet que cette période de stage et réalisé en priorité en zone sous-dense en fonction de l'offre de stage dans chaque région et des politiques d'incitation locales par une instruction interministérielle du 24 février 22, le gouvernement a initié une politique incitative de recrutement de maîtres de stage en zone sous-dense parce qu'il faut avoir les étudiants, mais il faut avoir aussi les maîtres de stage qui les accueille pour accroître ses torts Offres de stage et augmenter le nouveau, le nombre d'étudiants qui s'y engagent cette instruction rappelle que les stages ambulatoires doivent constituer une véritable opportunité pour les étudiants en médecine de découvrir des spécificités de l'exercice ambulatoire, elle rappelle aux ARS et aux universités que les multiples leviers existants pour développer et diversifier l'offre, l'offre dans les zones sous-denses, doivent être mobilisées dans tout leur potentiel, le gouvernement fixe des objectifs ambitieux de développement et de diversification de ses stages, nous voulons notamment accroître de 7 le 7 % % d'ici 2024 le nombre de maître de stage universitaire formé parce qu'il faut des formations là aussi des maîtres de stage sont ainsi être intégrés sont aussi intégrée au Plfss pour 2023 avec l'incitation à effectuer une nouvelle 4ème année de consolidation en fin d'internat de médecine générale en priorité dans les territoires Soudan.

je trouve qu'on va là encore une fois assez vite et puis je profite de de cet instant et de ses 30 secondes que je peux m'adresser à vous pour vous lance un SOS. Vous êtes ministre en charge des personnes handicapées, il y a une autre urgence aujourd'hui partout, on est en attente de place en IME, on est en attente de place des dates, on est en attente de prix que vous connaissez comme moi le pris acte de notre région, nouvelle Aquitaine plus de création de places pour personnes handicapées, plus de personnes, création de placer de lits en Ephad c'est une des conséquences des constats que l'on voit aujourd'hui dans les différents d'ailleurs rapports sénatoriaux, donc il y a vraiment une urgence et je vous remercie de l'entende ce matin, merci madame la présidente. Merci, cher collègue, la parole est à présent à monsieur Jean Michel Arnaud. La présidente, Madame le Ministre, mes chers collègues, ma question porte sur les conséquences des réseaux de soins fermé pour les professionnels et les patients, ces réseaux de soins mettent en relation les assurés avec les professionnels de santé et on joue un rôle dans le rapport qualité prix des prestations fait en baisser les prix, toutes ces années, a paru dans les années 90 il se sont développées au milieu des années 2000, avec le lancement de plateforme de gestion pour le compte d'organismes complémentaires d'assurance santé cependant la problématique actuelle provient de la loi dite Le Roux du 27 janvier 2014 qui est ces réseaux à pratiquer des remboursements différenciés, cela signifie que les mutuelles peuvent différencier leur prise en charge en toute légalité dans des domaines peu couvert par la Sécurité sociale dans l'optique l'odontologie, par exemple, en fonction des praticiens consultés ou des professionnels sollicités dans un rapport de 2017 l'IGAS précise que cette législation comporte des dispositions trop générale pour avoir une réelle portée et ont permis à ces réseaux de se développer dans un cadre essentiellement concurrentiel gaz dénonce également le fait que la relation contractuelle entre les plateformes et les professionnels de santé et elles-mêmes déséquilibré en plus d'être conclu sans aucune négociation, ces conventions comportent une très forte asymétrie des droits et obligations réciproques en définitive ces système de remboursement différencié son facteur d'inégalité d'inéquité pour les patients et d'injustice pour les professionnels, avec un service rendu de moindre qualité, la pression à la baisse des prix tel qui s'exercer au finalement non par ailleurs plus d'utilité depuis la mise en place de l'Ordre 100 % santé depuis le 1er janvier 2021, nous avons donc affaire à une forme d'américanisation, une partie de notre sécurité sociale, dont l'égalité l'universalité devraient être les valeurs cardinales, Madame la Ministre, quelles sont les intentions du gouvernement en vue de mieux encadrer ces pratiques en limitant notamment les effets néfastes pour les professionnels non mutualiste et surtout qu'est la position quand une potentielle suppression des dispositions prévues par la loi, l'Roux merci. Merci, cher collègue, pour vous répondre Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur Jean Michel Arnaud. Les réseaux de soins permettent de modérer les tarifs de soins et d'équipements de santé un rapport de l'IGAS de juin 2017 mettent en évidence, en effet, en observant un écart de prix notable entre les soins ou produits consommés via un réseau et se consommer au réseau, particulièrement dans le domaine de l'optique, moins 20 % pour des verres adultes moins 10 pour pour les montures les réseaux permettent également de modérer la progression des primes d'assurance complémentaire de plus depuis la réforme du 100 % % santé qui supprime les restes à charge dans l'optique, il ne peut plus y avoir de remboursement différencié que les équipements soient achetés dans un réseau ou non du point de vue des professionnels, le Conseil constitutionnel dans une décision de 2014 n'a pas estimé que les conditions d'adhésion aux réseaux de soins étaient de nature à porter une atteinte disproportionnée à leur liberté d'entreprendre, ces derniers sont libres d'adhérer au réseau ou non et peuvent le quitter à tout moment, enfin, le rapport de l'IGAS, observe que l'encadrement des offres permet d'accroître la lisibilité pour l'assurer, notamment dans le secteur de l'optique qui présente une multitude de produits plus de 50000 références de verre par exemple, l'asymétrie d'information entre professionnels et patients semble ainsi réduite tant du point de vue de l'assurer que de celui du professionnel de santé, le fonctionnement actuel des réseaux de soins ne semble pas devoir être réformé, mais le gouvernement restera vigilant et prendra des mesures si la situation venait à le justifier. Oui, Madame la Ministre, j'entends vos propos, je constate simplement, dans mon département, un certain nombre de préparation à l'accompagnement des usagers et des patients se fait dans chez des opticiens et qu'au bout du compte ses opticiens malgré le travail de préparation vont leur clientèle, leur échapper, ce qui n'est pas normal compte tenu des conditions tarifaires auxquels je j'ai fait allusion dans mon interrogation, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à présent notre collègue, Madame la sénatrice critique Herzog. La présidente, monsieur le Ministre, la situation déficitaire d'offre de soins et de formation de nouveaux médecins dans le département de la Moselle est alarmante, la désertification médicale est omniprésente, pourtant le département compte plus d'un 1000000 d'habitants, soit presque 50 % de la Lorraine, mais ne possède pas de centre hospitalier universitaire un CHU, les Mosellans doivent se rendre à Nancy, via l'autoroute A31 saturé en Meurthe-et-Moselle, département voisin de 731 habitants seulement cette étrangeté fait du département de la Moselle, le parent pauvre de la santé publique hospitalière avec une densité de 126 médecins pour 100000 habitants que la Meurthe-et-Moselle en compte 164 qui plus est, l'Agence Régionale de Santé l'ARS du Grand-Est basé à Nancy, a procédé à la suppression de 598 emploi et de la fermeture de 174 lits en 2020 pendant la pandémie l'Allemagne nous à leur reprocher le manque de lits pour les travailleurs frontaliers alors que sévissait le variant Sud-Africain très agressif, je me suis battu contre les décisions de l'Allemagne et et fait appel, le président de la République qui a pu obtenir de Berlin à la mi-mai 2021 un infléchissement des contraintes subies par les travailleurs frontaliers dans leur cour, ce qu'on les contres les tests des 48 heures au-delà de cet épisode très douloureux et se gare de de de nombreux patients décédés, la désertification de la médecine rurale en Moselle, m'amène à vous demander de créer urgemment un centre hospitalier universitaire pour Parlier à notre retard si je salue la volonté du gouvernement d'affecter les internes en quatrième année dans dans les zones sous-dotées en pratique ambulatoire, encore faut-il en avoir un, les étudiants ne viendront pas de Nancy, il est évident que le CHU, Metz, Thionville permettra la dotation de la terre de 4ème année en stage de pratique ambulatoire surtout départements au bénéfice de nos patients ce CHU et demandée par la population, les soignants, les dirigeants, les élus et les patients, il est urgent, Monsieur le Ministre, que vous nous fassiez part de votre de Merci, chers collègues, je confie à Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées vous répondre. Merci madame la présidente, madame la sénatrice Christine Herzog C H R U de Nancy honte initié depuis plusieurs années une dynamique de rapprochement devant notamment permettre l'univers si starisation du 1er dès 2009 des premiers échanges ont permis la mise en oeuvre d'une communauté hospitalière de territoire de convention d'associations ont été signés en 2011 et 2014 cet enjeu a connu une avancée décisive en 2019 avec une 3ème convention associant également l'ARS grande test cet accord décide lettrés, de ce qui pourra devenir un grand ensemble hospitalo-universitaire lorrain dans la mise en oeuvre de cette convention, il était prévu que 5 services soient identifiés pour élaborer un projet médico- universitaire à date un consensus existe pour l'hématologie l'odontologie, la pharmacie et les urgences, le choix du 5ème service n'a pas encore été tranchée si la mise en oeuvre de la convention a été impacté par la crise Covid les travaux ont repris en 2021 les discussions menées non pas pour le moment, permis aux 2 établissements de se mettre d'accord sur les orientations et les objectifs à atteindre aussi une mission conjointe de l'IGAS et de l'inspection générale de l'Éducation du sport et de la recherche sera lancé dès novembre, elle fera le point sur la démarche engagée identifiera les difficultés et proposera des orientations sur cette démarche d'université Ariza Sion, dont la pertinence a été réaffirmée par la directrice générale de l'ARS et la présidente de l'Université de Lorraine je vous promets. Merci, la parole est à présent à notre collègue sénateur Monsieur Hervé Maurey pour poser sa question orale. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, depuis mon élection au Sénat, la question des déserts médicaux est au coeur de mon action car elle constitue un sujet majeur pour nos territoires ruraux convaincu que seuls les mesures incitatives ne suffiront pas à mettre un terme à une situation de plus en plus préoccupante je propose depuis près de 15 ans une régulation à l'installation des médecins comme elle se pratique dans un certain nombre de pays et comme nous la pratiquons nous même pour un certain nombre de professionnels de santé, les gouvernements successifs s'y sont toujours refusés pourtant, chacun peut constater que les mesures mises en place depuis plus de 20 ans sont insuffisantes, puisque la situation ne fait que se dégrader après un quinquennat de déni, la question des déserts médicaux n'avait même pas été identifiés dans le cadre du grand débat, le candidat Emmanuel Macron s'est prononcé le 17 mars dernier pour le conventionnement sélectif, je le cite ce vers quoi je souhaite qu'on avance, c'est de stopper les conventionnement dans les zones qu'on considère comme bien doté, c'est un mécanisme qui est efficace, je n'aurais pas dit mieux cet engagement se retrouve également à la page 9 de son programme, toutefois depuis la réaction de prendre la République cet engagement semble avoir disparu, il n'est plus question que de prévention qui, si elle est utile et nécessaire n'est pas suffisante pour régler ce problème, pas plus que le ne le serait la quatrième année d'internat professionnalisante aujourd'hui envisager je souhaiterais donc savoir, Madame la Ministre, si le gouvernement souhaite oui ou non mettre en oeuvre les engagements du président de la République sur ce sujet ou s'il entend y renoncer. Merci pour vous répondent Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur. Auteur l'accès aux soins et à la santé est une priorité gouvernementale forte dès 2017, le plan d'accès aux soins, a mis en place une large palette de solutions comme le soutien à la réalisation des stages ambulatoires, le développement des maisons et centres de santé pluri-professionnelles ou la création des communautés professionnelles territoriales de santé, l'enjeu, sachant que les bénéfices de la suppression du du numerus clausus ne se feront pas sentir avant quelques années, et de continuer à mobiliser tous les leviers existants pour libérer du temps médical et augmenter l'attractivité des territoires comme la facilitation des consultations avancées ou encore la télémédecine la stratégie ma santé 2022 a permis la création de 4000 postes d'assistants médicaux pour seconder et appuyer les médecins, libérant ainsi pour eux du temps médical le Ségur de la santé, a renforcé le déploiement de l'exercice coordonné et le recours à la télé, santé, les réponses sont à chercher sur le terrain, dans une logique de différenciation et de responsabilité partagée et le volet santé du Conseil national de la refondation va permettre de mettre autour de la table, les professionnels, les patients, les élus de chaque bassin de santé afin de trouver les réponses les plus adaptées aux besoins spécifiques des populations en parallèle déchanter nationaux sont accélérés comme pour les assistants médicaux dont la cible a été porté à 10000 à l'horizon 2025 les communautés professionnelles territoriales de santé, les femmes C devront couvrir l'ensemble du territoire d'ici 2023 et se mobiliser prioritairement sur l'accès au médecin traitant les dispositions ambitieuses sont aussi intégrée au Plfss pour 2023, notamment l'incitation à effectuer l'année de consolidation en en médecine générale en priorité dans les territoires sous-denses qui n'a pas l'air de vous convaincre, mais qui peut être une solution pour ben bien faire connaître les territoires aux étudiants mais. Merci, cher collègue, vous avez une poignée de secondes, si vous souhaitez répliquer. Ma question était très simple est-ce que le gouvernement va mettre en place l'engagement d'Emmanuel Macron, pendant la campagne présidentielle de mettre en place un conventionnement sélectif pour l'installation des médecins, vous ne m'avez pas répondu, vous avez rappelé ce qui avait été fait par le gouvernement précédent et qui, malheureusement, les faits sont là et les chiffres le montrent est insuffisant, donc je considère que cette non-réponse vaut sans doute renoncement à la promesse du président de la République pendant sa campagne, je le regrette et je vous donne, Madame la Ministre, rendez vous à la fin de ce quinquennat et où, malheureusement, nous constaterons à nouveau une dégradation de la situation en matière de démographie médicale, je le regrette. La parole est à présent un autre collègue sénateur Monsieur Georges Patient. Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, Madame la Ministre, la situation de la production d'électricité et très critique en Guyane, le taux de disponibilité électrique s'il est connu et certainement catastrophique car toutes les communes de Guyane, sans exception aucune, sont confrontés à des coupures intestins intempestives longue, trop souvent, en plus des déficits dépistage programmé plusieurs se raisons à cela : la trop grande vétusté des installations le sous-dimensionnement du réseau et des moyens de production, mais aussi et surtout les lenteurs administratives qui viennent freiner, voire bloquer leur remplacement, je vais vous citer de cas concrets, début octobre, la commune de Maripasoula déjà enclavé, a connu plusieurs jours de Blackout total suite à la panne simultanée de ces 4 générateurs, avec pour conséquence directe, l'absence d'eau potable de téléphone les écoles fermées, pourtant concernant cette commune, il existe de projet d'unités de production électrique, inscrit dans la programmation plus pluriannuelle de l'énergie depuis 2017, il devait être mis en service en 2021 le soir entier en 2023 autres autre cas, la centrale thermique de dégrader qui assure 30 à 40 % de la production électrique du territoire pour être remplacé avant fin 2023, et de façon impérative, elle doit être remplacée par la centrale du Larivot à chantier à l'arrêt suite à des recours, les travaux devraient reprendre, mais pour quelle date de mise en production, que va-t-il se passer en 2000 madame la Ministre, le président de la République a récemment affirmé à Saint-Nazaire sa volonté d'accélérer, d'aller 2 fois plus vite dans le déploiement des énergies renouvelables, la Guyane eurent et gare aux retards accumulés devra bénéficier d'un rythme encore plus grand si on veut qu'elles sortent vraiment de cette insécurité énergétique criante. Merci, cher collègue, pas vous répondre, j'invite Madame Bérangère Couillard, secrétaire d'État chargée de l'écologie au micro. Merci madame la présidente, ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs les les sénateurs, monsieur le le sénateur patient vous avez interrogé madame Agnès Pannier-Runacher Ministre de la Transition énergétique, nous pouvons être présente, elle m'a chargé de de vous répondre, la production d'électricité en Guyane, fait l'objet d'une attention toute particulière, l'état et la collectivité de Guyane ont acté le remplacement de la centrale de de grade des cannes par une centrale située à Larivot, fonctionnant au bio-liquide les travaux de construction ont été arrêtés en raison de de plusieurs contentieux le 11 octobre 2022, à la suite de la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux, de suspendre l'exécution de l'annulation du permis de construire, le ministre de la transition énergétique et des mer ont demandé à EDF de reprendre les travaux pour une mise en service fin 2026, cela nécessite une prolongation de la centrale de de grade des cannes jusqu'à cette date, aujourd'hui l'essentiel de la production est assurée par le barrage de petits la priorité est donnée aux installations de production basées sur le photovoltaïque et la biomasse, bien que vieillissante, la centrale de de grade, assure l'équilibre offre-demande au quotidien avec 2 moteurs déclassé et de en maintenance sur ces 9 moteur des turbines à combustion assure le secours la spatialisation actuel des moyens de production impose pour une bonne résilience du système électrique des projets, notamment dans l'ouest guyanais, le projet si E G a malheureusement pris du retard. Dans les communes de l'intérieur non interconnectées, la production et surtout assurée par des centrales thermiques vieillissantes, même si de nombreux projets de production décarbonés émerge comme à Saint-Georges à Maripasoula une série d'avaries, a récemment touché plusieurs moteurs est fortement perturbé la fourniture d'électricité qui est redevenu nominal une centrale photovoltaïque devrait entrer en service en 2024 et les travaux sur le projet de barrage bien d'autres comme le prévoit le code de l'énergie, la programmation pluriannuelle de l'énergie, co-élaboré par l'État et la communauté territoriale de Guyane, elle doit être révisée, des groupes de travail se sont réunis depuis mai pour définir les grandes orientations sur l'autonomie énergétique en 2030, il convient de souligner que la production d'électricité sera quasiment entièrement renouvelables à cette échéance, elle représente un peu plus d'un tiers de la consommation d'énergie finale en Guyane contre 62 % pour les transports. Merci madame la ministre, je voudrais saluer le conseil municipal des enfants de l'Aisne ans dans le Finistère à l'Inde, invitation de notre sénatrice Madame merci de votre visite. Je passe la parole à présent à notre collègue sénateur Jean-Pierre Corbisez. Merci monsieur le président de c'est vrai qu'il un peu chaud qu'on pourra peut-être montrer l'exemple en baissant un peu le thermostat, Madame la Ministre, mes chers collègues, le dispositif 0 artificialisation nette inscrit dans la loi climat et résilience inquiète fortement les élus locaux, je l'ai déjà dit ainsi dans mon département, à l'occasion d'échanges avec des maires ou des présidents d'intercommunalités ont été sauvé les points suivants d'abord l'articulation complexe, voire impossible, entre l'impératif Dusan les engagements d'une commune, dotée d'un programme ANRU nécessitant de bâtir avant de détruire, deuxièmement la problématique des communes rurales, confrontées à des difficultés réelles pour obtenir des friches à reconquérir pourtant essentiels à leur avenir, troisièmement la nécessaire prise en compte du phénomène du recul du trait de côte, les calculs Dusan afin de ne pas pénaliser davantage les communes du littoral me semble donc nécessaire d'avoir une implication Dusan différenciées et adaptées aux différents territoires et leur spécificité, et en particulier d'abord de tenir compte des efforts déjà consentis dans la réduction des consommations foncière comme dans le traitement des friches industrielles ou militaires d'exclure du décompte d'filiation, les projets d'intérêt national, voire supranationales telles que canal Seine Nord ou le réseau Express Grand Lille qui pénalise ces collectivités dans leurs projets de développement, de mettre en place des mécanismes correcteurs et de solidarité à l'échelle nationale ou régionale pour permettre d'accompagner la réalisation des projets structurants, en particulier dans les zones rurales ou littorales, je vais donc savoir, Madame la Ministre, quelles mesures le gouvernement dans le cas de sa volonté affichée d'agir en concertation avec les acteurs concernés, entend mettre en oeuvre pour corriger ses impacts. Merci, chers collègues, je voudrais vous témoigner par ma voix que nous appliquons la sobriété énergétique au palais, la preuve, j'invite Madame Bérangère Couillard, secrétaire d'État chargée de l'écologie à vous répondre. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les les sénateurs, monsieur le sénateur Corvisier, la mise en oeuvre du Dusan est crucial pour préserver la qualité de nos sols, la biodiversité, permettre un aménagement durable de nos territoires et combattre des effets du changement climatique autre son discours au XVIIIe congrès des régions de France à Vichy, la première ministre a confirmé cet objectif pour 2050, ainsi que l'étape intermédiaire prévue en 2031 d'une division par 2 du rythme de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, la loi 3DS avait déjà permis un report de 6 mois des échéances prévues par la loi climat et résilience ainsi les Scott ont jusqu'au 22 octobre pour se réunir et faire leurs propositions aux régions les régions disposent également de 6 mois de plus pour intégrer les objectifs de la loi climat dans leur sera dette soit jusqu'au 22 février 2000 vingt-quatre ce calendrier laisse donc un délai de mise en compatibilité significatif pour initier cette réforme est essentielle, cette ambition réaffirmée : le gouvernement est naturellement à l'écoute des élus locaux et du Parlement et il y a engagé depuis plusieurs mois, des concertations pour anticiper cette transformation majeure pour nos territoires le gouvernement tient à réaffirmer ici aujourd'hui que la trajectoire de réduction de l'artificialisation prendra en compte de nombreux critères afin de s'adapter aux singularités des territoires à leur projet à leur histoire, ainsi que le prévoit d'ailleurs la loi, la mise en oeuvre, Dusan dans les territoires doit également passer par un accompagnement des élus locaux pour favoriser les efforts de renaturation et de traitement des friches, c'est par exemple l'objet du Fonds friche qui a mobilisé 700 750 millions d'euros sur la période 2021 2022 au service de plus de 1118 projets pour réhabiliter, plus de 2700 hectares de friches, le fond d'accélération de la transition écologique contribuera à cette politique, à partir de 2023 doté de plus de 2 milliards d'euros, il permettra de financer des projets d'adaptation des territoires au changement climatique dont la renaturation des villes et le recyclage des friches dans nos territoires. Merci madame la ministre, chers collègues, vous avez une poignée de secondes pour. Oui, une solution existe le Ministre pour que les communes rurales récupère le foncier à bâtir en douane zones agricoles, c'est la PPL notre ancien collègue sénateur, ministre Jacques Mézard sur la procédure d'expropriation des biens en état manifeste d'abandon voter ici au Sénat, intégré dans la loi DS est aujourd'hui applicable et permet ainsi de réduire de 20 ans à 10 ans, les délais de récupération de sourcils malheureusement aujourd'hui, il n'existe pas de ligne budgétaire spécifique pour que ces opérations communal puisse se faire, il faudra peut-être effectivement que le gouvernement puisse y penser. Merci, Merci, cher collègue, la parole est à présent à notre collègue sénateur Monsieur Frédéric Marchand. Merci madame la présidente, madame la Ministre, je voudrais attirer votre attention et celle du gouvernement sur le sujet de l'indemnisation pour frais de déplacement des élus, l'ancien maire de drinks quand et ancien président de l'Association des maires ruraux du nord Luc m'a m'a en effet interpellé au sujet de l'indemnisation des élus qui représentent leur père dans leur cadre des commissions départementales, convoquée par le préfet, la commission départementale de coopération intercommunale, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, la commission départementale d'aménagement commercial pour n'en citer que quelques-unes sont bien évidemment nécessaires au bon fonctionnement de nos territoires et au-delà de notre démocratie, or les maires des communes modestes et celles éloigner de la préfecture, hésitent à s'impliquer dans ces commissions, car elles ont un coût en matière de déplacements et de temps à consacrer cela a souvent pour conséquence que ces commissions dont la composition est censé représenter l'ensemble du département se résume finalement à la réunion d'élus proches géographiquement du chef-lieu de département où se déroulent les dix de commission essentiellement pour éviter le coût du déplacement et un coup temps conséquent cette sous-représentation des territoires éloignés de la préfecture dans les commissions est une réalité dans le département du Nord, et on peut aussi l'a constaté dans l'ensemble des départements français pour y remédier, il serait utile de proposer un remboursement par l'état de ses frais de déplacement dont bénéficieraient les élus représentants leur père dans ces commissions, en effet, dans ce cas de figure l'élu n'agit pas pour l'intérêt de sa commune, auquel cas des fragments est prévu mais pour l'ensemble des élus du département ce défraiement par l'État permettrait que ces commissions soit réellement représentatif de l'ensemble du territoire départemental, par ailleurs, le financement de ce défraiement pourraient être imputés sur la dotation générale de fonctionnement et le coût serait neutre pour les finances de l'état aussi, je vous remercie de m'indiquer quelles mesures financières peuvent être prises afin que les élus éloignées du chef-lieu départemental puissent être défrayés pour leur participation aux commissions départementales et ainsi représentées équitablement le territoire départemental merci. Merci, cher collègue, la parole est à Bérangère Couillard, secrétaire d'État chargée de l'écologie. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les les sénateurs, monsieur le sénateur Marchand le gouvernement n'ignore pas les difficultés que peuvent rencontrer les élus locaux qui consacrent leur temps et mettent leurs compétences au service de leur territoire, leur rôle au sein des différentes commissions départementales convoquée par le préfet est à cet égard particulièrement central en participant à ces organes consultatifs il il assure la représentation des collectivités territoriales du département dans différents champs de politiques publiques qui relève en tout ou partie de la compétence de l'État, afin de garantir le bon fonctionnement de ces instances de proximité et la représentation de l'ensemble des intérêts concernés, le décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État consacre la prise en charge des frais de déplacement pour les personnes qui prennent part à des organismes consultatifs conformément à l'article 2 du décret précité et concerner toute personne qui se déplace pour, je cite, participer aux commissions conseils comités et autres organismes consultatifs dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics, les commissions départementales sont présidées par le préfet et leur organisation relève de l'État qui prend en charge leur secrétariat et leurs frais de fonctionnement, l'article 2 du décret permet ainsi d'inclure les élus qui se rendent aux réunions de commissions départementales instaurée par l'État, ceux-ci sont donc éligibles au remboursement de leurs frais de transport, sur la même base forfaitaire que celles applicables aux fonctionnaires civils de l'État, le gouvernement est particulièrement vigilants au bon fonctionnement de ces instances qui participent au travail commun entre l'État et les territoires. Merci, cher collègue, vous avez 6 secondes pour répliquer parfait je donne donc la parole maintenant à notre collègue sénatrice Madame Viviane Artigalas. Merci madame la présidente, madame la Ministre, premier plan majeur pour les territoires de montagne depuis 40 ans, le plan à venir montagne investissement financé par l'État avec six régions à 331 millions d'euros au massifs français pour leur permettre d'adapter leur économie qui dépend en grande partie de la saison hivernale, de s'adapter aux mutations du tourisme et d'assurer leur transition écologique, plusieurs pistes sont envisagées : rénovation de l'immobilier et actions sur les lits froids, développement d'un tourisme Vert et 4 saisons, révision de la chaîne des mobilités et des services entre vallées et stations d'altitude pour le seul massif des Pyrénées : ce plan permettra de Mumbai mobilisé 54 millions d'euros pour financer des projets de transition touristique, 2 questions se posent cependant l'adaptation locale de la mise en oeuvre du plan, les élus craignant une année inadéquation entre les investissements annoncés et l'effectivité réelle de leur réalisation sur le terrain, l'autre question concerne la pérennisation de ce plan et des montants alloués car les crédits court jusqu'en fin 2022 il faudrait a minima, prévoir une extension à 2023, des capacités de programmation afin de de pouvoir accompagner de nouveaux projets d'intérêt pour la transition touristique qui n'ont pas pu être faute de crédits suffisants par ailleurs il fraudé et tendre de 2 ans supplémentaires, la période d'appui du plan à venir montagne January actuellement limitée à 2 ans, ce qui est trop court pour réaliser les projets des territoires sélectionnés, madame la ministre, pouvez-vous nous confirmer que ce dispositif sera bien maintenu, je vous remercie. Merci, cher collègue, Bérangère Couillard secrétaire d'art, chargée de l'écologie, pardon, va vous répondre. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Artigalas le plan à venir montagne lancé par le 1er ministre le 27 mai 2021 est aujourd'hui bien avancé et connaît les réalisations suivantes, les 150 millions d'euros d'investissements apportés par l'État sur 2021 2022 seront engagés en totalité d'ici cette fin d'année au profit de projets d'investissements, porté par les territoires en 2021 140 projets d'investissements ont été accompagnés à hauteur de 50 millions d'euros, et en 2022 près de 300 projets d'investissements seront accompagnés à hauteur de 100 millions d'euros complémentaire au titre du volet ingénierie le PAM prévoit par ailleurs trois enveloppes d'ingénierie en soutien aux territoires de montagne 62 territoire bénéficie d'un accompagnement vers un modèle touristique plus durable est résiliant via le financement d'un chef de projet, l'accès à une offre de services déployés par une vingtaine de partenaires et d'une animation dédié correspondant à la mobilisation de 10 millions d'euros de l'État et 6 millions d'euros de la banque des territoires sur 2021 2022 10 millions d'euros auront également été mobilisés d'ici fin 2022 en faveur de la mobilité du 1er et du dernier kilomètre dans les territoires de montagne une seconde vague de lauréats viendra en octobre s'ajouter aux 58 lauréat, déjà désigné au printemps 2022, enfin 5 millions d'euros sont seront mobilisés par la banque des territoires et atout France au profit de la rénovation de l'immobilier de loisirs sur 25 stations lauréate dans une optique de réflexion sur le logement et le tourisme afin de mesurer les plans, les effets du plan montagne et de mieux cerner les problématiques qui doivent encore être traités dans ces territoires. Ma collègue Dominique Faure, secrétaire d'État chargé de la ruralité, va prochainement faire une tournée des massifs afin de rencontrer, associations, acteurs économiques, et bien sûr les élus autour de la définition de leur besoin en ingénierie et en investissements dans les 2 années à venir, cette tournée des massifs sera complété par l'organisation d'une concertation nationale visant à identifier les besoins sur d'autres thématiques. Merci madame la Ministre, il vous reste 29 secondes pour répliquer. Merci, oui je le ce, ce plan à venir montagne a été saluée par tous les élus de la montagne, particulièrement par la même, mais je crois qu'il est important de continuer le travail sur ce sujet vous annoncer des choses, mais c'est vrai que les élus ont besoin vraiment que ce plan soit soit poursuivi au-delà des échéances, initialement annoncé pour lui permettre de produire ses plein un effet et, plus largement, les territoires et les acteurs, ces territoires de montagne en ont besoin et on vous remercie de continuer à y attacher une intention soutenu merci beaucoup. Merci, la parole est à présent à notre collègue sénateur, monsieur Jacques Fernique. derniers tronçons des lignes 17 nord et 18 ouest du Grand Paris Express et de la gare du triangle de Gonesse, à première vue, ces projets paraissent vertueux, selon la cour d'appel de Paris la ligne 17 nord s'inscrit dans la stratégie de report modal, que nous appelons de nos voeux, constitue une alternative à la voiture et contribue donc à préserver l'environnement, car ne répondant pas, ne répondant pas aux besoins des habitants actuels, elle ne trouveraient leur justification qu'au travers d'une urbanisation massive des Terres agricoles, présenté comme un nouvel axe majeur pour le nord de Paris, la ligne 17, ses 26 kilomètres et demi de ligne 9 gares et 13 communes concernées à l'origine, elle avait été proposée, on s'en rappelle, dans le cadre du projet pharaonique EuropaCity heureusement abandonné cet abandon aurait dû logiquement entraîner l'arrêt des travaux au de la de la gare du Bourget, aéroport et ceux de la gare triangle de Gonesse, dont les bénéfices sont très limités, le projet ne va en rien profiter aux habitants des communes alentour, trop éloigné, sa rentabilité et même discuté l'aéroport Roissy Charles de Gaulle constitue aujourd'hui une barrière à l'urbanisation son franchissement au nord, mettrait en péril l'existence des Terres seine et marnaise et picarde des Terres agricoles parmi les plus riches d'Europe, où est la volonté de freiner l'étalement urbain en 2018, un rapport de la Cour des comptes à demander au gouvernement de revoir le calendrier, le périmètre du projet, ce dernier n'a pourtant jamais été modifiée en novembre 2019 le TA de Montreuil avait estimé l'étude d'impact et les mesures compensatoires la Société du Grand Paris, juge et partie, à la fois n'a pourtant jamais revu sa copie, ma question est donc double : dans quelle mesure le gouvernement entend poursuive le développement du tronçon contesté de la ligne 17 la réalisation de la gare triangle de Gonesse, ainsi que la ligne 18 au-delà de Saclay, le gouvernement va-t-il étudier la possibilité d'un moratoire sur ces différents projets pour engager une étude d'impact indépendante. Merci, cher collègue, pour vous répondre Madame Bérangère Couillard, secrétaire d'État chargée de l'écologie. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les les sénateurs, monsieur le le sénateur faire nique la ligne 17 nord du Grand Paris Express doit favoriser le développement des territoires entre Paris et Roissy l'abandon du projet EuropaCity ne remet pas en cause la création de la gare triangle de Gonesse situés entre les aéroports du Bourget et de Roissy et à proximité de la zone d'activité de Paris-Nord, elle est la seule gare du Grand Paris Express implantée dans le département du Val-d Oise, les dessertes de cette gare et les interconnexions faciliteront l'accès des habitants du département au bassin d'emploi, les projets autour de cette gare ont évolué et les emprises sont maintenant réduite pour chacun de ces projets, c'est un développement économique sur la transition agroécologique et l'agriculture urbaine qui est visé, je citerai le projet Agora Lim, portée par la C. Maris que vous soutenez ou encore la filière agricole de la future Cité scolaire internationale. Enfin, le Conseil d'État a rejeté le 17 octobre le pourvoi formé par plusieurs associations, il a ainsi validé l'autorisation de création et d'exploitation de la ligne 17 accordées en 2018 cela conforte le projet, dont les travaux sont déjà bien avancés, le tronçon ouest de la ligne 18 constituent la colonne vertébrale transport du projet scientifique, technologique et urbain, porté par le l'Établissement public d'aménagement de Paris-Saclay dans le cadre d'une opération d'intérêt national, il ne peut être mis en cause pour sans porter atteinte au projet et aux synergies déjà engagée et menée en concertation avec l'ensemble des acteurs, le projet du Grand Paris Express va contribuer au désenclavement de territoires aujourd'hui peu ou mal desservies au bénéfice des Franciliens et du développement régional. Merci, la parole est à présent à notre collègue Jean-Claude Tissot. Merci madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, la nécessaire transition en cours dans le secteur des mobilités avec la décarbonation progressive de nos modes de déplacement implique de nombreux enjeux et axes d'évolution ainsi l'aménagement de nos territoires donc dorénavant prendre en compte l'électrification des véhicules et, logiquement, prévoir les infrastructures adaptées et cette volonté d'accompagner le développement des véhicules électriques s'est concrétisé dans plusieurs dispositions législatives en effet l'article 118 de la loi climat et résilience indique que les parcs de stationnement de plus de 20 emplacements gérée en délégation de service public en régie ou via un marché public dispose d'au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables

plusieurs collectivités de mon département, interpellés et de la communauté de communes Charles humainement plus récemment et confrontée à ces difficultés pour l'ensemble de ces parcs de stationnement, monsieur le Madame le Ministre, pardon, pouvez-vous nous préciser les modalités exactes de ces obligations ainsi que les principaux éléments de calendrier, est ce que l'ensemble des parkings publics de plus de 20 place jouxtant ou non un bâtiment public sont concernés par les obligations est ce que ce dispositif concerne uniquement les projets à venir où l'ensemble des parcs de stationnement déjà construit dans ce sens serait-il possible de nous préciser la notion de parcs de stationnement évoqué dans cet article est-ce que les parkings publics publics de stationnement libre ont les mêmes obligations que les parkings payants, il est également évoquée dans le texte de loi que la répartition des bornes de recharge peut s'effectuer sur plusieurs parcs de stationnement d'un territoire donné est-ce que cette répartition logistique et financière peut être penser à l'échelle intercommunale. Enfin, le questionnement du financement de ces installations, inquiète également fortement les collectivités comme souvent l'État annonce de belles dispositions qui doivent finalement être portés par les collectivités, sans aucun Zenga engage sans aucun accompagnement face à de nouvelles charges dans des Budgets déjà déjà particulièrement limitée sur ce dispositif, l'accompagnement de l'État est indispensable, pouvez-vous nous indiquer si le gouvernement, qu'on ne prend des engagements pour accompagner financièrement et logistiquement les les collectivités territoriales à ce sujet est-ce que le fond Vert annoncé par Madame la première ministre pourrait participer à ce soutien financier, je vous remercie madame. Merci, cher collègue, la parole est à Madame Bérangère Couillard, secrétaire d'État chargée de l'écologie, je ne sais pas si vous aurez assez de temps pour répondre à toutes ces questions. Je vais tenter, madame la présidente, mesdames et messieurs les les sénateurs, monsieur le sénateur Tissot pour atteindre la neutralité carbone en 2050 l'état engage résolument la transition vers les véhicules électriques nécessitant l'installation de bornes de recharge l'homme donne ainsi la possibilité aux EPCI organisatrice autorités organisatrices de mobilité et autorité organisatrice de distribution d'électricité, de réaliser des schémas directeurs de développement des infrastructures de recharge, ouverte au public, facultatif, ce dispositif donne à la collectivité, un rôle de chef d'orchestre du développement de l'offre de recharge sur son territoire, il vise à aboutir à une offre coordonnée entre les maîtres d'ouvrage publics et privés, cohérente avec les politiques locales de mobilité et adaptée aux besoins, la loi climat et résilience français schéma obligatoire dans les ZFU FM pour accompagner ces collectivités dans la réalisation de ces schémas, l'État a publié un guide méthodologique et met à leur disposition plusieurs jeux de données en Open Data, par ailleurs, la banque des territoires pourra être mobilisée sur l'élaboration d'un schéma directeur, lorsque celle-ci s'appuie sur un prestataire externe là l'homme prévoit en outre que jusqu'à fin 2025 le raccordement au réseau public de distribution d'électricité des s'inscrivant dans un schéma directeur peut être pris en charge jusqu'à 75 %, un arrêté ministériel en cours de finalisation définira les modalités précises d'application l'homme porte également dans le code de la construction et de l'habitation, l'obligation d'équiper dès 2025, d'un point de recharge par tranches de 20 places les parkings de tous les bâtiments non résidentiels, qu'il soit privé ou public, dans le cadre de la loi climat résilience des collectivités ont une obligation assez similaire d'équiper d'un point de recharge par tranches de 20 places et d'ici 2025 les parcs de stationnement en délégation de service public en régie ou gérés par un marché public, le gouvernement a renforcé les mesures de soutien au déploiement de ses infrastructures de recharge ainsi le programme de certificats d'économie d'énergie à devenir visant à aider financièrement les collectivités dans le déploiement de bornes à la demande a été abondée début 2022 de 200 millions d'euros et prolongé jusqu'en 2025 les territoires ont d'ores et déjà activement mobilisées ce programme et en complément, le gouvernement a annoncé dans le cadre de France 2030, une enveloppe de 300 millions d'euros pour des appels à projets de déploiement de stations de recharge à haute puissance. Merci, la parole est à présent à notre collègue Madame Céline Brulin. Merci madame la présidente, madame la ministre, alors que la nouvelle ligne Paris-Normandie n'en finit plus de se faire attendre le seul TGV normand est menacée, la SNCF a en effet annoncé une inversion des horaires de la ligne qui dessert Le Havre, Rouen, Lyon et Marseille et à partir du mois de décembre, le TGV partirait du Havre vers Marseille, en milieu d'après-midi et, inversement, le matin de Marseille pour rejoindre le à vers 14 heures 30 sept un non-sens au regard des usages, car cela ne correspond absolument pas aux besoins des voyageurs de cette ligne transversale qui permet d'éviter un changement à Paris et c'est évidemment précieux, c'est un non-sens pour toute la Normandie, puisque ce changement d'horaire pacte aurait bien évidemment les correspondances comme celle de Caen, Dieppe ou encore Cherbourg c'est enfin un non-sens qui fait l'unanimité contre lui, en témoigne l'adresse commune que l'ensemble des parlementaires de Seine-Maritime a adressé au directeur général de la SNCF à travers laquelle nous lui demandons de revoir sa copie, ce qui se joue en fait, c'est l'avenir de cette desserte, car la décision de la SNCF à rendre cette ligne moins attractive est-ce que c'est pour justifier de la supprimer dans quelques temps ce n'est pas parce que sa compétence est circonscrite aux trains d'équilibre du territoire que l'État doit se désintéresser des dessertes TGV encore moins dans une région si peu investi par les lignes à grande vitesse et qui a déjà perdu une ligne TGV, celle qui faisait Le Havre Strasbourg il y a quelques années maintenant et donc ma question c'est : quelles sont les démarches que le gouvernement entend mener aux côtés des élus que nous sommes pour contraindre la SNCF à garantir des horaires adaptés pour le TGV Le Havre-Marseille je vous remercie. Merci, cher collègue Madame Bérangère Couillard, secrétaire d'État chargée de l'écologie pour vous répondre. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice brûle, le gouvernement est attentif à ce que l'offre de transport ferroviaire, soit en mesure de répondre aux besoins de mobilité dans les territoires, à ce titre, la loi de 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire prévoit la mise en place depuis fin 2020, d'une information obligatoire de l'État et des collectivités territoriales, par les entreprises opérant des services librement organiser lorsque celle-ci souhaite les modifier et et ce afin d'anticiper les difficultés éventuelles, vous l'avez précisé, Madame la sénatrice, la SNCF a ainsi annoncé à l'État et aux collectivités concernées le repositionnement horaires de sa liaison TGV entre Marseille et Le Havre à partir de décembre 2022, avec un départ du Havre à 15

d'une part l'optimisation de sa production, et en particulier de la gestion de sa maintenance et, d'autre part, l'amélioration du remplissage de ces trains qui est aujourd'hui limitée, l'enjeu n'est donc pas de fragiliser mais bien de redonner une dynamique à cette ligne qui peinent encore à trouver son public, j'entends les interrogations des élus et les usagers qui ne partagent pas la même appréciation de l'opportunité de ces évolutions, le gouvernement invite la SNCF à faire preuve de plus de pédagogie pour expliquer la motivation de son projet et dissiper j'espère les inquiétudes en tout état de cause, il sera utile que la SNCF tire un bilan de l'exploitation de ce service, avec un recul de quelques mois et puis s'en partager les résultats avec les élus, plus largement, le développement de nouvelles lignes transversales relève avant tout de choix stratégiques de la SNCF et d'autres entreprises ferroviaires en fonction de leur évolution du marché en ce qui concerne les lignes susceptibles d'être conventionnée par l'État, les travaux qui avait été menée en 2021, dans le cadre de l'étude remise au Parlement sur les perspectives de développement de nouvelles lignes de trains d'équilibre du territoire n'pas conduit à identifier de potentielles suffisant pour des lignes au départ de la Normandie dans ce cadre. Merci, cher collègue, il vous reste quelques secondes pour répliquer. Je suis un peu inquiète, Madame la Ministre parce que redynamiser une ligne comme vous dites que la SNCF entend le faire en choisissant des horaires qui sont à l'heure actuelle renier enfin refusé par les usagers, c'est évidemment le contraire de ce qu'il faut faire et je crains que, ils ne suffisent pas, de faire de la pédagogie, je crois qu'il faut faire faut avoir des mesures qui rendent cette ligne attractive, elle est utile pour relier de grands ports que sont Le Havre et Marseille, et je crois que vous devriez être à nos côtés pour exiger qu'elle demeure en l'état. R collègue, la parole est à présent à notre collègue le sénateur Max Brisson. Merci madame la présidente, madame la Ministre, les trains de nuit ont un bilan carbone 15 fois moins important que l'avion et propose un coût unitaire par passager largement inférieur au TGV et constitue donc de véritables atouts pour la politique de mobilité nationale en alliant à la fois vertus écologiques et valorisation du transport ferroviaire, voilà pourquoi le gouvernement a rétabli de lignes de trains de nuit au départ de Paris, l'une pour Nice, l'autre pour Tarbes, via Limoges et Toulouse et c'est ici que le bât blesse car la SNCF a fait le choix d'une desserte de Sud-Ouest par l'itinéraire défini en 2011 via Toulouse, elle a abandonné le tracé initial qui, à partir de Dax reliés en 2 rames, Bayonne, Hendaye, Irun, d'une part et Pau, Lourdes, Tarbes, d'autre part, elle la remplacer par un itinéraire via Toulouse ne t'es Servent Pau, Bayonne et Hendaye que l'été, dans des conditions dégradées, c'est d'ailleurs ce trajet qui avait provoqué en 2011, une augmentation du temps de transport, une baisse de la fréquentation et finalement la suppression de la ligne, ce choix n'est donc pas le bon, c'est réduire le sud des Landes et les pénates Atlantique à une desserte uniquement estivale alors qu'il ne peut être séduit réduits à de simples territoires touristiques, ce sont des pôle économique dynamique et des foyers de population conséquent qui mérite une desserte cohérente et faciliter, Madame la Ministre, quelles sont les raisons précises qui ont privilégié le jeu, le choix d'un tracé il y à Limoges et Toulouse, seriez-vous prêt à rétablir une liaison régulière par train de nuit suivant l'axe Atlantique historique via Bordeaux, celui qui assure la meilleure desserte des Landes et du Pays basque, du Béarn et de la Bigorre. Si cher collègue, madame la secrétaire d'État, je vous invite à répondre à notre scène. Madame, madame la présidente, pardon je vous avais pas madame la présidente, merci messieurs dames et messieurs les les sénateurs, monsieur le le sénateur Brisson je partage votre conviction que les trains de nuit, on a un avenir, en effet, il constitue une offre de transport écologique et sociale alors qu'il ne restait plus qu'en 2020 que 2 lignes de nuit l'étude transmise au Parlement en mai 2021 conformément à la loi d'orientation sur les mobilités donne des perspectives de renouveau de ce mode de transport déjà dans le cadre du plan de relance de lignes ont été ouvertes en 2021 Paris-Nice et Paris-Tarbes et Aurillac devrait être desservis en décembre 2023 130 millions d'euros seront investis dans la rénovation du matériel et des installations de service, dont 100 millions d'euros de France relance des décisions doivent être prochainement prises sur la consistance du futur réseau de trains de nuit, le renouvellement du matériel roulant, les modalités de financement avec une perspective d'ouverture à la concurrence de l'exploitation d'ici quelques années, la desserte du Sud-Ouest par train de nuit fait partie de cette problématique et devra être pensé dans ce cadre plus général aujourd'hui la nécessité la nécessaire régénération de l'infrastructure ne permet pas des horaires optimaux et limite la desserte à Tarbes et Lourdes en dehors de l'été dans les prochaines années, il faudra également organiser la desserte en prenant en compte les travaux dans les noeuds de Bordeaux et de Toulouse, je peux déjà vous indiquer qu'à partir de 2000 vingt-quatre le train de nuit desservira quotidiennement Dax, Bayonne, Orthez et Pau, en plus de Lourdes et de Tarbes, ces évolutions positives montrent tout l'engagement de l'État en faveur de ce mode de transport pratique et respectueux de l'environnement. Merci Charles Max vous avez quelques secondes. C'est à la présidente donc si j'ai bien compris en 2024 vous respecterez la promesse du président Bacrot qui avait déclaré la palombe bleue, je l'ai pris plein de fois, il faudrait investir ici, donc si vous avez bien entendu matin Ministre c'est bien par Bordeaux et Dax, que le train de nuit passera pour desservir le Béarn et le Pays basque, cité les le cas, ce serait une avancée, j'espère que cette réponse se concrétisera en 2024. Merci, la parole est à présent notre collègue sénateur monsieur Stéphane Demilly. Merci madame la présidente bonjour madame la Ministre, l'augmentation des des prix de l'énergie est aujourd'hui la première source d'inquiétude de nos concitoyens, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures pour tenter de répondre à la situation dramatique qui se profile, cet hiver, c'est bien et je ne rentrerai pas dans le débat de savoir si c'est suffisant ou pas, je souhaite néanmoins de façon non polémique vous alerter sur 2 sujets spécifiques tout d'abord celui des granulés de bois, en effet, vous le savez, dans beaucoup de foyers de nos concitoyens, ils ont installé des poêles et chaudières à bois, bénéficiant ainsi de primes environnementale mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, il n'est pas certain qu'il puisse acheter des granulés de bois d'une part à cause de l'inflation exponentielle de ces matières et, d'autre part, tout simplement parce qu'il n'aura peut être plus sur le marché pour l'hiver 2022 en France, ce sont environ 850000 foyers qui sont équipés d'un chauffage au Pelé ou granulés de bois face à cette situation, des mesures autres que le chèque énergie sont-elles envisagées pour ce type particulier de chauffage, telle est le 1er point de ma demande 2ème sujet qui concerne spécifiquement mon mon département plus exactement ma ma région, celui des endiviers, confrontés à des hausses de coûts de l'énergie, présenté par les opérateurs pouvant attendent jusqu'à plus 800 vous avez bien entendu plus 800 % l'énergie est déjà un poste très important du prix de revient des endives du fait des caractéristiques calorifique nécessaire dans une salle de forçage pour faire pousser l'endive, ces entreprises sont donc aujourd'hui clairement en péril, or le dispositif d'aide, gaz, électricité, mise en place par le gouvernement ne permet pas de répondre aux spécificités de chaque filière, avez-vous été saisi de ce problème et qu'envisagez-vous de faire pour ce secteur économique très prégnant dans les Hauts-de-France, j'ai naturellement bien sûr alerté votre collègue en charge de l'agriculture pour qu'ils viennent, le cas échéant nous rencontrer sur place. Merci, cher collègue, la parole est à Bérangère Couillard, secrétaire d'État chargée de l'écologie. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les les sénateurs, monsieur le sénateur, vous vous le savez, nous faisons face à la plus grave crise énergétique depuis les chocs pétroliers de de 1970 la guerre en Ukraine et de est venue accentuer le coût des matières premières et du transport, cela aussi impacté le prix des granulés de bois en parallèle de la hausse des prix de l'électricité, du gaz et du fioul, on assiste à la constitution de stocks prudentielles qui accroît la pression sur la demande pour ces raisons des distributeurs ont pu faire face à des ruptures de stock temporaire face à cette situation, le gouvernement agit pour répondre à la disponibilité des granulés à court et long terme et pour soutenir financièrement les Français qui subissent la hausse des prix tout d'abord, les producteurs et distributeurs de granulés travaillent à assurer l'approvisionnement en granulé des consommateurs français, cet hiver, le ministère de la transition énergétique a aussi mis en place dans le cadre de France 2030, des mesures qui permettront d'augmenter les capacités de séchage des produits bois et donc de production de granulés, c'est notamment le cas de l'appel à projets si Beitia tu bois chaleur Industrie Agriculture et tertiaire, l'Ademe à contribuer au financement de 14 chaufferie lié à à la fabrication de granulés, ce qui représente une production annuelle de granulés, estimé à 850000 tonnes concernant les aides aux ménages et notamment les plus modestes, un chèque énergie exceptionnel de 100 euros avaient été 10 attribué à 5 8 millions de ménages en décembre 2021 ce chèque est utilisable jusqu'au 31 mars 2023 et permet de régler des factures d'électricité, de gaz de fioul ou d'autres combustibles dont notamment le bois un nouveau chèque énergie exceptionnel sera envoyé à 12 millions de ménages en fin d'année, soit 40 % des ménages de 200 euros pour les 5 8 millions de ménages les plus modestes et 100 euros pour les autres, s'agissant des aides aux entreprises, je veux vous réaffirmer le soutien du gouvernement aux entreprises : nous ne laisserons pas tomber dans les entreprises, les TPE sont déjà protégés par les bouclier tarifaire, vous avez cité le ai le guichet résilience dont nous avons élargi les critères pour qu'ils bénéficient à plus d'entreprise il y a également la R N H qui a permis d'éviter une hausse d'au moins 60 % de leur facture aux entreprises, énergie, le gouvernement a décidé d'aller plus loin dans cette protection, c'est pourquoi un amendement sera déposé au PLF. Pour prévoir un mécanisme de garantie, dont les modalités seront précisées dans les prochains jours, monsieur le sénateur, je tiens à vous assurer de la mobilisation totale du gouvernement pour accompagner les Français et les entreprises à faire face à la crise énergétique, j'en profite, mesdames et messieurs les sénateurs, pour vous remercier pour l'attention que vous m'avez porté tout au long de ces questions qui étaient sur les sujets de transition écologique énergétique et je souhaite, madame la présidente, un prompt rétablissement. Merci Bérangère la parole, vous avez une poignée de secondes pour Merci madame la présidente, madame la ministre, bien que répondant au souhait de création de commune nouvelle regroupant plusieurs communes historique, les élus locaux subissent le refus de la Poste d'attribuer un code postal unique la la commune nouvelle ainsi créée, au moment où la simplification est un objectif affiché par tous, une commune nouvelle se voit conserver plusieurs codes postaux source évidente d'erreur d'adressage mais se voit confronté également à l'impossibilité de répondre aux demandes de ses administrés d'une certification d'adresse postale, les sites internet de l'État et de la Poste étant en contradiction je souhaiterais donc savoir, Madame la Ministre, si des mesures simples et de bon sens ne pourrait pas être initié et prise afin que la Poste harmonie sur un même territoire un code postal unique au nom de la commune nouvelle la mention de la commune, déléguée pouvant apparaître dans le corps de l'adresse comme un lieu-dit et ceci évitant la problématique des homonymes de voix des homonymie de voix, je vous remercie. Merci, cher collègue a bienvenue Madame Caroline Cayeux, ministre délégué chargé des collectivités territoriales. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur, c'est pour limiter les difficultés liées à l'adressage dans les communes nouvelles que les anciens codes postaux ont été maintenus, ce qui permet à la Poste de garantir la distribution du courrier, si je suis persuadé, derrière ça va être compliqué, l'attribution des codes postaux dépend exclusivement de la Poste et de son organisation, des bureaux distributeurs à chaque bureau distributeur est associé un code postal distincts et les communes avec plusieurs bureaux distributeurs ont de ce fait plusieurs codes postaux, cette pratique ne concerne pas que les communes nouvelles, mais également les grandes communes ou celle avec des aspérités géographique, si je comprends les difficultés que vous soulevez je ne peut que relever que l'harmonisation des codes postaux d'une même commune qui est possible, en théorie, s'il existe un centre de tri unique et après une concertation approfondie a parfois conduit à des perturbations dans l'organisation du tri postal, j'ajoute que l'impossibilité de voir une adresse reconnue sur des plateformes Internet n'est pas lié au code postal, mais à la nécessité de mettre l'adresse à jour au sein de la base adresse nationale l'article 169 de la loi 3DS reconnaît pleinement la compétence de la commune en matière d'adresse, le conseil municipal étant chargé des dénominations de voix et des lieux-dits de leur numérotation après insertion des adresses dans la banane, La Poste se charge de leur fiabilisation qui estime que seulement 8000 communes ont procédé à une certification au moins partielle de leurs adresses, je vous invite donc là où se posent des difficultés que vous soulevez monsieur le sénateur, à encourager les maires à actualiser les adresses de la commune. Merci, cher collègue, il vous reste quelques secondes. et des mères ce problème de code postal est un réel problème et on a du mal à faire entendre raison à La Poste, dont le devoir d'accompagnement en termes d'aménagement du territoire devrait être une des premières missions, me semble-t-il, d'une telle société. là, pardon, la question est à présent à notre collègue sénateur Jean Raymond et Gonnet. Merci madame la présidente, madame la Ministre, chers collègues depuis de trop nombreuses années, le phénomène des constructions illégales est devenue un véritable fléau pour nos communes, l'absence d'un réel traitement administratif et juridique efficace renforcent dangereusement le sentiment du 2 poids, 2 mesures auprès de nos concitoyens, or depuis quelques temps maintenant une nouvelle étape vient d'être franchie dans mon département, l'Essonne, plus de 60 pour 100 des communes sont confrontées à la prolifération de constructions illégales inhérentes au détournement de droit de préemption urbain par le biais de la signature d'un bail emphytéotique. Les malfaisants font usage d'une faille juridique, révélé par la jurisprudence de la Cour de cassation qui a jugé, dans une décision du 11 mai 2000 que le droit de préemption urbain s'applique à des mutations de propriété mais non à des mutations de jouissance, cette faille permet de contourner le droit de préemption, rien de plus simple, il suffit de signer un bail emphytéotique bail qui peut être, je le rappelle, d'une durée de 99 ans, et qui permet de devenir quasi propriétaire à moindre prix, sitôt le terrain loué des constructions bafouant les règles d'urbanisme en vigueur sortent de terre au nez et à la barbe du maire et des riverains, les maires ont alors pour seul recours, le dépôt de plainte aujourd'hui, ce sont des centaines de procédures interminables et sans effets qui sont en cours dans le département, nous sommes là devant un détournement manifeste de la réglementation, il est plus qu'urgent de faire cesser ce phénomène dévastateur, quelles mesures comptez-vous prendre, Madame la Ministre, pour y parvenir. Merci, cher collègue, la réponse est donc à Madame Caroline Cayeux Ministre délégué chargé des collectivités territoriales. Merci madame la présidente, monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, Hugonnet comme vous l'avez dit, le 11 mai 2000, la Cour de cassation a jugé que le bail à construction ainsi que le bail emphytéotique ne sont pas soumis au droit de préemption urbain toutefois si le contrat de bail prévoient que la propriété du bien loué doit être transféré aux preneurs en fin de contrat, la cession à titre onéreux des droits réels immobiliers tels que le droit réel immobiliers conférée par un bail emphytéotique ou à construction est soumise au droit de préemption urbain, cette décision est transposable au droit de préemption en espace naturel sensible en l'état actuel de la réglementation, la déclaration d'intention d'aliéner s'applique uniquement à des mutations à titre onéreux, donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrain, le juge rappelle cependant que si le bail emphytéotique prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du bail, ce dernier sera lui, soumis au droit de préemption dans les espaces naturels sensibles par ailleurs les règles en matière de construction et d'aménagement de coupes et abattages d'arbres ou de stationnement de caravanes sont très restrictives en zone naturelle et en zone agricole, le refus d'autorisation en matière de droit des sols en conformité avec les règles d'urbanisme dont la compétence appartient au maire de le PCI, selon le cas est également de nature à favoriser la protection de ces espaces sensibles et à les préserver, il appartiendra donc au notaire chargé d'établir le bail de déterminer si ce dernier est soumis au droit de préemption en espace naturel sensible selon l'effectivité du transfert de la propriété, à la date d'expiration du bail, il est recommandé à l'ensemble de la profession, représentée par le Conseil supérieur du notariat, la plus grande vigilance sur ce point. Merci madame la ministre, et il vous reste 25 secondes Chers collègues pour répliquer. C'est plus qu'il n'en faut, madame la présidente, je vous remercie madame la midi je sais que pour avoir été mères que vous êtes parfaitement consciente du sujet, vous nous vous nous avez rappelé le droit que nous connaissons par coeur, en revanche, et mon collègue maire de longs ponts sur Orge Alain l'amour qui est dans la tribune. C'est pour montrer le fossé qui existe entre la réalité sur le terrain et ce qui se passe en réalité, c'est-à-dire un maire face à un problème sur lequel le droit ne va pas au bout des choses, il est urgent, urgent, Madame la Ministre, que nous, nous nous en parlions de ce sujet, merci de votre attention. Merci, chers collègues, avant de vous donner la parole, cher collègue, Cathy ah pour ce police je voudrais saluer la très nombreuses délégations qui vous accompagne avec les enfants de la commune de Vimy, merci de de votre visite, collègue, à vous la parole pour votre question orale. Merci madame la présidente, madame la ministre, permettez-moi, madame la ministre d'avoir une pensée particulière pour les habitants des village de Bihucourt en cours Les Cagnicourt Bucquoy Ervillers Maury et ceux et celles victimes de la tornade de ce dimanche, certains ont tout perdu, je salue ici les maires élus, pompiers, gendarmes et services de l'État et du département, les agents d'Enedis et tout ce sur le pont depuis dimanche soir, au côté du ministre Darmanin nous avons pu constater hier l'ampleur des dégâts le 14 octobre dernier nous avons organisé, madame, dans le Pas-de-Calais, un rassemblement porté par plusieurs dizaines d'élus maires d'élus face aux dépenses des collectivités qui explose, les collectivités territoriales réalise 70 % des investissements publics essentiels à nos populations aujourd'hui des projets sont remis en cause au vu des prix des énergies, des matériaux, des denrées alimentaires qui flambent, les maires doivent choisir quel service ils suspendent pour leur population, il protège à travers les CCAS, les populations qui font face à des difficultés croissantes le bouclier tarifaire ne s'appliquera pas à l'ensemble des communes, la hausse de la DGF de temps 320 millions d'euros est insuffisante, nous demandons qu'elle soit indexé sur l'inflation 2023 et qu'il y ait une augmentation madame la Ministre de 770 millions d'euros pour le bloc donc qui peut faire face à l'inflation de 2023, madame la ministre, il faut que le gouvernement étende y compris le bouclier tarifaire à toutes les communes, sans distinction de taille, qu'en pensez-vous je vous remercie. Eh bien, nous allons le savoir avec la réponse de Madame Caroline Cayeux Ministre délégué chargé des collectivités territoriales. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Cathy ah pour Sow avant de vous apporter ma réponse, je voudrais vous dire qu'à mon tour je partage aussi vos propos de soutien aux communes dévastées, hier et avant-hier et je tiens à vous assurer, évidemment, de tout notre soutien à ces communes dont j'ai eu certains maires au téléphone hier alors sur la question que vous me posez, le gouvernement est pleinement conscient des effets de l'inflation sur la situation financière des collectivités territoriales et agit en conséquence, il a en lien avec le Parlement, mis en place un ensemble de mesures permettant d'apporter les premiers éléments de réponse aux collectivités territoriales, je voudrais vous rappeler le bouclier tarifaire qui a été adoptée pour limiter à 4 % en 2000 22 et à 15 % en 2023 la hausse des dépenses d'électricité des communes de moins de 10 agents dont les recettes sont inférieures à 2 millions d'euros et ce dispositif pourrait concerner, d'après nos calculs, près de 28000 communes en 2ème lieu la loi de finances rectificative d'août dernier, a institué ce filet de sécurité pour accompagner budgétairement les communes et leurs groupements, le coût du dispositif est estimé à 430 millions d'euros et les collectivités pourront jusqu'au 15 novembre sollicité un acompte sur ce montant, avant la fin de l'année 2022, le gouvernement propose de reconduire un dispositif de même nature, centré sur les dépenses énergétiques au titre de l'année 2023 dans le cadre des débats sur le projet de loi de finances en 3ème lieu pour la première fois depuis 13 ans, le gouvernement a décidé d'augmenter de 320 millions d'euros la DGF en 2023 ce soutien concret notifié au 1er trimestre 2023 devrait permettre à plus de 90 pour 100 des communes de voir leur DGF progressé ou tout au moins être stabilisée par rapport à l'année 2022 l'ensemble de ces mesures qui vont être précisées dans le cadre du débat parlementaire autour du projet de loi de finances 2023 montre que le gouvernement est aux côtés des collectivités pour leur permettre de faire face aux défis de l'inflation. Si Madame la Ministre, vous avez une poignée de secondes, chers collègues, pour répliquer. Merci, ça va, ça va tenir, madame la ministre, les maires demandent quand même quelles garanties auront-t-il sur la compte de 2023 2 DGF versé en 2022 donc je vous demande d'être particulièrement vigilante et il y aura-t-il des reprises de DGF l'an prochain en cas de trop-perçu parce qu'actuellement, ils n'ont pas beaucoup de visibilité, je vous remercie. Merci, chers collègues, je voudrais saluer le conseil municipal des jeunes de Saint-Julien les villas, nous avons beaucoup de visite aujourd'hui à l'invitation de Madame Evelyne Perrot, sénatrice de l'Aube, merci de de votre visite, cher collègue Monsieur Yves Détraigne, la parole est à vous, monsieur le sénateur. Merci madame la présidente, madame la ministre, depuis que j'ai déposé cette question orale en août, le ministre de l'Intérieur a eu l'amabilité de répondre au courrier que je lui avais également adressé le même jour sur le sujet n'y voyait pas une forme de harcèlement de ma part mais plutôt la volonté d'obtenir une réponse pour mémoire ces interventions venez après 3 questions écrites et un courrier resté tous sans suite, pourtant, la question est simple : jusqu'à quel moment une municipalité doit pouvoir prendre en compte une procuration de vote dématérialisé, la circulaire du 24 mai 2022 indique qu'on ne peut pas refuser une procuration au peu au motif qu'elle est tardive et recommande, dans la mesure du possible aux mairies de tenir une permanence, cela ne veut pas, ça ne peut pas satisfaire les est-ce élus communaux soit le ministère ordonne de tenir une permanence et en fixe les horaires soit-il, il impose un délai clair pour en finir avec les procurations de dernière minute, monsieur Darmanin dans sa réponse du 2 septembre dernier qu'on vient des difficultés techniques et pratiques engendrés par la dématérialisation des procurations et précise qu'il faudrait fixer en concertation avec les associations d'élus, une date limite pour l'établissement de ces documents, je vous demande donc aujourd'hui quand le cadre juridique sera mis en adéquation avec la réalité des contraintes de nos communes. Merci, cher collègue, Madame la ministre Madame Caroline Cayeux, ministre délégué chargé des collectivités territoriales pour vous répondre. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur, Yves Détraigne, aucun, aucune disposition du code électoral n'impose de date limite pour établir une procuration de vote qui peut donc en théorie être établi le jour même du scrutin, nous connaissons les difficultés qu'engendre cette absence de date butoir, notamment le risque que les procurations tardive ne puisse pas être pris en compte par les communes du fait des délais d'acheminement postaux, l'introduction des procurations dématérialisé dont je souligne qu'elles sont plébiscitées par les électeurs, puisqu'elle représente 69 % des 3 7 millions de procuration de procuration établie en 2022, et je dirais qu'elles amplifient ces difficultés puisqu'elle donne aux électeurs un faux sentiment d'immédiateté en outre la gestion centralisée des procurations dans le répertoire local électoral unique depuis le 1er janvier 2022 qui allège la charge des communes implique que les contrôles de validité effectué par celle-ci se fasse au moyen d'un poste informatique alors dans ce contexte, il a été recommandé aux communes de mettre en place, dans la mesure du possible des permanences le jour du scrutin pour vérifier les procurations tardive, j'ai conscience que cela a pu conduire à mettre sous tension, certaines communes qui ont pu rencontrer des difficultés pour y procéder, c'est pour cette raison qu'à l'issue du bilan des élections législatives et présidentielles, nous examinerons en étroite concertation avec les associations représentées représentatives des collectivités territoriales, les modalités d'introduction d'une date limite pour l'établissement des procurations afin de mettre le cadre juridique en adéquation avec la réalité des contraintes vécues par les communes. Si Madame la Ministre, la parole est à présent à notre collègue, Madame la sénatrice, Laurence Cohen. Merci madame la présidente, madame la ministre ma question porte sur la situation des travailleurs sans-papiers de l'agence Chronopost à Alfortville, ces hommes intérimaire employé essentiellement sur des des postes de tri et de manutention sont en grève depuis décembre 2021, l'une des plus grandes grèves longues, en tout cas dans ce secteur, ils se mobilisent aux côtés d'organisations syndicales d'élus pour obtenir leur régularisation et faire respecter leurs droits, malgré plusieurs demandes, la direction du groupe La Poste, dont Chronopost est une filiale, refuse de remplir le Cerfa de régularisation de plus, il semblerait qu'il y a un contournement contournement organisé et volontaire de la circulaire Valls aujourd'hui comme lors du conflit précédent de 2019 La Poste société à capitaux publics à cent pour cent dont 34 % détenus par l'État ne reconnaît pas ses responsabilités d'employeur et se réfugie derrière ses sous-traitants, Madame la Ministre, quand l'état va-t-il prendre ses responsabilités en régularisant au plus vite ces salariés qui constituent une main-d'oeuvre corvéable à merci, quand allez-vous avec le ministre du Travail, mettre un terme au scandale de la sous-traitance en cascade au non respect du code du travail à ce système d'exploitation des travailleurs les plus précaires par l'État lui-même. Merci, cher collègue, Madame la Ministre, je vous invite à répondre à notre collègue sénatrice. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Laurence Cohen, vous m'interrogez sur la situation notamment au regard du droit de au séjour des travailleurs sans-papiers de l'agence Chronopost d'Alfortville, je sais que ces salariés en situation irrégulière sont en grève depuis plusieurs mois maintenant, en réaction à des conditions de travail qu'ils estiment difficiles et à une mobilisation jugée insuffisante de leur employeur pour entreprendre les démarches nécessaires à leur régularisation si les dépôts groupée de demande de régularisation sont une pratique courante dans le cas de conflits sociaux, je voudrais vous rappeler que la décision d'admettre à titre exceptionnel à l'individu au séjour relève du préfet du département de résidence de chacun des étrangers qui statue individuellement sur chaque demande le droit au séjour, je voulais vous rappeler, c'est un droit individuel la régularisation prend en effet en compte le niveau d'intégration dans la société française et d'adhésion aux valeurs de la République et ne peut intervenir si l'étranger constitue une menace à l'ordre public, la procédure d'admission à titre exceptionnel, nécessite de transmettre à la préfecture compétente plusieurs documents pour chaque salarié concerné, dont un Cerfa complétée et signée par l'employeur. Sachez que les préfets de la région d'Île-de-France ont été sensibilisés sur ce dossier et vont examiner les demandes transmises selon ses orientations, enfin, s'agissant du non respect du code du travail, c'est à la justice éclairée par les constats effectués par l'inspection du travail et les investigations qu'elle est susceptible de diligenter qu'il appartient d'apprécier et de qualifier cette situation complexe et de déterminer la responsabilité des différentes parties prenantes. Merci, cher collègue, il vous reste 45 secondes pour parler. Oui, merci, Madame la Ministre, je connaissais le mode d'emploi de la régularisation, le problème qui vous est soumis aujourd'hui, c'est que ce sont des travailleurs qui sont exploités par la Poste et par les sous-traitants, que vous le savez, que l'État le sait et quand vous parlez d'intégration dans la société, quelle est la meilleure intégration que de travailler comme ils le font et sont ce qu'on respecte leur parole parce qu'ils sont obligés de décharger des camions que la cadence est infernale et d'ailleurs, Madame la Ministre, je voudrais dire que pendant la crise du Covid ils ont continué à travailler et que ça a permis à la Poste de faire plus de 45 de d'augmentation d'activité sans que ça ruisselle sur les salariés, donc il faut arrêter l'hypocrisie, il faut absolument qu'ils soient régularisés, il y a les travailleurs de RSI, qui l'ont été suite à une lutte, il faut que aussi soient régularisés, il faut arrêter la sous-traitance en cascade, qui est un véritable scandale, une pratique de surexploitation et il y a la responsabilité de l'État qui est complètement engagé dans ce processus, donc c'est le sens de ma demande et j'espère que suite à cette question orale et à toutes les mobilisations qui qui mobilise de nombreux élus, hé bien vous allez enfin entendre leur leur voix parce que on ne peut pas les considérer en 2022 comme de véritables esclaves qui n'ont absolument aucun droit, je vous remercie madame. Collègue, la parole est à présent un autre collègue sénateur Monsieur Michel Savin. Merci madame la présidente, madame la Ministre, en 2008, la France a instauré un moratoire sur l'utilisation des machines à voter depuis, seul un petit nombre de communes est autorisé à utiliser ces appareils l'homologation de nouveaux modèles et donc interdites comme votre collègue ministre de l'Intérieur, l'a reconnu le moratoire en vigueur est devenue une source de risques Alain Pichon, les communes de renouveler leurs machines dans de bonnes conditions, en effet, face au manque de débouché commercial, les producteurs ont cessé de fabriquer les machines à voter homologué les communes autorisées continue donc d'utiliser leurs vieux appareils ces mêmes communes seront particulièrement confronté au problème de l'ouverture de nouveaux bureaux de vote lorsque leur population augmente en octobre 2018, la commission des lois du Sénat a publié un rapport sur le vote électronique, préconisant de mettre fin au moratoire de 2008, ma question est double : madame la Ministre votre collègue ministre de l'Intérieur a demandé il y a 18 mois à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, d'engager une étude de sécurité nécessaires à la sortie du moratoire, quelle est la position du gouvernement après cette étude à l'écart du moratoire et quelques quelles réponses comptez-vous apporter aux communes qui utilisent des machines à voter et qui doivent équiper de nouveaux bureaux de vote. Merci, cher collègue, Madame la Ministre, je vous engage à répondre. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Michel Savin, les machines à voter sont prévues en droit français depuis 1969 et des modèles électroniques sont autorisés depuis 2003, toutefois le périmètre des communes autorisées à en être équipé ainsi qu'à acquérir de nouveaux modèles et gelé depuis le moratoire de 2008, du ministre de l'Intérieur, les services du ministère de l'intérieur en lien avec l'Anssi Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques ont donc, comme vous l'avez dit engagé une réflexion pour réaliser examiner le cadre applicable aux machines à voter et les et l'évolution technique requise en vue d'une éventuelle levée du moratoire dans cette perspective, le gouvernement a remis au Parlement le 17 décembre 2021, un rapport sur la possibilité de recourir aux machines à voter conformément à la loi du 22 février 2021, ce rapport inclut les résultats des travaux réalisés en coopération avec Lancy les travaux engagés se sont appuyés sur une démonstration de machines à voter, actuel, un échange avec des homologues belges seul utilisateurs en Europe à ce jour de machines à voter, ils ont vu et et fait aussi une analyse de risques et des études techniques et c'est ce rapport qui précise les conditions dans lesquelles le statu quo pourrait être levé au terme de ce rapport, la levée du statu quo et maintenant subordonnée à des modifications substantielles des modèles de machines à voter autorisé et de leur processus d'homologation et ces modifications incluent notamment l'impression d'un bulletin papier pour rendre le vote par machines à voter, vérifiable et Audi table voilà les réponses que je voulais vous apportez si chers collègues, vous avez 45 secondes pour répliquer. M. la présidente, madame la ministre, votre réponse et et partiel : aujourd'hui les communes qui se retrouvent dans ses difficultés attendent une autre réponse du gouvernement, soit il y a une possibilité de continuer à maintenir les machines à voter, au niveau des communes et il faut leur donner la possibilité de pouvoir, soit trouver des machines anciennes qui puisse s'adapter aux machines qui sont déjà d'actualité sur ces communes soient cette ce dispositif pour arrêter les machines à voter, mais il faut que la position soit claire on ne peut pas continuer à accepter que dans certaines communes communier des machines à voter, et sur d'autres bureaux de vote, on ne puisse pas équiper ses bureaux de vote de machines à voter, qui crée des tensions et des disques et des et un mode de fond en fonctionnement qui est différent selon les bureaux de vote, la même commune, donc nous ce qu'on attend à ce qu'attendent ces communes-là, c'est une réponse claire du gouvernement, j'ai bien entendu que ce rapport a été remis qu'aujourd'hui des modifications doivent apporter, il faut que rapidement ces communes soient informés sur sur ces nouveaux dispositifs. Merci, la parole est à présent à notre collègue Jean Marie misons. Merci madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, notre République repose sur des principes intangibles, le respect de la loi en éteint et puisque nul n'est censé ignorer la loi, nous devrions tous avoir à l'esprit que selon l'article 16 du code de procédure pénale, le maire 1er magistrat de sa commune est officier de police judiciaire, il peut donc constater des infractions et requis requérir le concours des forces de l'ordre à l'heure actuelle, le mépris de cette règle qui constitue déjà en soi un délit remet gravement en cause la légitimité de ses élus à intervenir dès lors qu'il constate des violations du droit c'est vraiment particulier chez les plus jeunes et de façon plus aiguë, parfois en zone rurale, à titre d'exemple, le maire de Timon ville en Moselle, confronté à de multiples manquements à la loi d'un adolescent de 16 ans est d'abord intervenu auprès de l'impétrant, sans succès, et puis à signaler les faits à la gendarmerie et enfin dresser procès-verbal des longtemps restée sans effet dans ces conditions, madame Ministre ne pensez-vous pas qu'une politique de sanctions plus sévères de ce type de comportement qui doivent systématiquement être l'objet de poursuites pénales doivent être mises en place, car l'exemplarité des peines encourues vous toute publicité sur les prérogatives d'maire merci. sur les prérogatives d'maire merci. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, Mison le gouvernement partage l'objectif de développer une réponse pénale efficace dans le cadre d'une action coordonnée entre les élus et l'autorité judiciaire, des efforts ont récemment été déployés en ce sens pour consolider les moyens juridiques et matériels mis à la disposition des élus municipaux pour faire appliquer leurs décisions, la loi du 27 décembre 2019 relatives à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique dites actions engagement et proximité à renforcer l'autorité, l'efficacité des mesures de police du maire, notamment par la création de nouvelles possibilités de sanctions administratives sous la forme d'amende d'un montant maximal de 500 euros, le cas échéant, après mise en demeure et astreintes le maire a donc désormais la possibilité d'infliger des sanctions administratives en cas de méconnaissance de ces arrêtés de police pour lutter contre certaines incivilités au quotidien, quand tu les actes portent atteinte à la sécurité des personnes et présente un caractère répétitif et connu, en outre, en application de la même loi, le procureur de la République est tenu d'informer le maire sur les suites judiciaires des infractions signalées et des plaintes déposées, qui le concerne, ou concerne sa commune, par ailleurs, la circulaire de politique pénale du garde des Sceaux, du 20 septembre 2022 a réaffirmé la nécessité d'un renforcement des relations entre les parquets et les maires, cet objectif est ainsi identifié comme l'un des éléments permettant le développement d'une justice de proximité favorisant la révélation des infractions commises, comme la mise en oeuvre des réponses individualisées graduée pour réparer le préjudice et éviter les récidives. Merci madame le ministre, il vous reste 45 secondes chers collègues si vous souhaitez répliquer. Merci madame la ministre, vous savez, le constat que je fais au travers de cette question, il peut être fait par tout à chacun, et en dépit des efforts que vous avez rappelé la situation ne change pas on peut le déplorer et quantité de mer sont découragés de voir que rien ne change, en dépit de texte adopté ici et à l'Assemblée nationale, il me semble que là qui fait défaut, c'est la rapidité avec laquelle la justice se saisit d'une affaire étrange cette affaire tant qu'on n'aura pas donné les moyens suffisants à la justice, combien même auront aura-t-on donner de nouveaux moyens à la police à la gendarmerie, on n'avancera pas suffisamment sur ce sujet, alors je forme le voeu, et puis si vous me reporté mon message auprès de qui de droit pour que les choses évoluent en ce sens, merci. Merci, cher collègue, la parole est à présent au sénateur Didier Rambaud pour sa question orale. compte tenu de votre engagement politique, y compris dans un département, l'Oise, que nous avons en partage et pour lequel nous souhaitons le meilleur, vous connaissez le sentiment d'abandon qui anime toujours plus d'habitants des territoires ruraux, il peut prendre plusieurs formes, la semaine dernière d'ailleurs, le Sénat a adopté une proposition de loi de Bruno Retailleau, que j'ai soutenu pour lutter contre le fléau que représente la désertification médicale mais aujourd'hui j'évoquerai le simple accès pour déposer une demande de renouvellement ou de délivrance des petites d'identité, carte et passeport car si la loi oblige à démontrer son identité comme on s'y soumettre, s'il faut attendre plusieurs mois, et faire de nombreux kilomètres pour déposer un dossier si les raisons de cet engorgement peuvent être conjoncturel, la crise sanitaire ayant retardé de nombreux concitoyens renouveler leur document, elles ne peuvent l'expliquer à elle seule, et si je peux entendre les motivations qui ont sous-tendu à la réforme de 2017, notamment pour mieux sécuriser ses titres la pratique révèle une fois encore, une rupture d'égalité manifeste au détriment de ceux qui habitent à la campagne, conscient de cette problématique, le gouvernement a lancé un plan d'urgence le 4 mai dernier dont je ne doute pas que vous allez nous en rappelé les grandes lignes, la loi de finances rectificative adoptée par le Parlement, a également prévu des mesures de soutien financier aux communes mais les 31 communes de l'Oise poseront des terminaux nécessaires ne peuvent absorber tout ce flux et les difficultés persistent, de nombreux maires relayons leurs administrés l'évoque lors de nos rencontre chaque semaine à cet égard, permettez-moi de vous rappeler que les maires aspirent notamment un allégement des normes à une visibilité sur l'évolution de la ressource, un meilleur fonctionnement des intercommunalités, ou encore à une amélioration de leur statut, Madame la Ministre, pour de nombreux concitoyens cette problématique est une preuve supplémentaire qu'ils sont des citoyens de seconde zone, des progrès sont à noter, je pense aux maisons de France service à condition que cela soit amplifiée, mais il vous faut obtenir des résultats et je sais pouvoir compter, comme les habitants du Beauvaisis sur votre volontarisme en la matière, je vous remercie. Merci madame la ministre madame Caroline Cayeux. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, Édouard Courtial, je vous rappellerai que dès 2018 l'État renforcer son accompagnement financier en revalorisant la dotation pour les Kids sécurisé versée aux communes dans lesquelles sont installés ces dispositifs de recueil en 2022 en face de la l'augmentation exceptionnelle des demandes de titres d'identité, le ministère de l'Intérieur a décidé d'un plan d'urgence pour accélérer le déploiement de nouveaux dispositifs de recueil et réduire les délais aujourd'hui anormalement long, j'en conviens avec une enveloppe de 14 millions d'euros adopté dans le PLFR d'août dernier, la dotation a été augmenté et rendu plus hein 17 y'incitative pour les dispositifs mis en place et pour les nouveaux dispositifs installés à titre pérenne ou temporaire, avec par exemple une prime de 4000 euros versés en plus des 4000 euros déjà prévus pour tout nouveau dispositif installé une trentaine de centres temporaires d'accueil équipé de 5 à 10 dispositifs de recueil temporaires ont donc été mis en place sur l'ensemble du territoire et cela correspond à l'installation de 221 stations de recueil supplémentaires au 1er juillet 2022, 4650 dispositifs de recueil, répartis sur 2464 communes sont désormais en fonctionnement, et comme vous l'avez dit, pour une plus grande proximité avec les usagers, de nouveaux dispositifs sont également déployés dans les espaces France services gérés par des mairies qui n'en disposaient pas dans ce cas, ce sont 183 communes qui ont été identifiés dès le printemps, et 74 on dort, j'ai déjà fait part de leur intérêt pour accueillir ce service, le réseau a donc été augmenté de manière pérenne de 10 % et les résultats sont là, les rendez-vous ont augmenté et dans le cadre de plans d'actions qui doivent permettre de réduire les délais de délivrance des titres d'identité, il est prévu de déployer 500 nouveaux dispositifs, notamment dans les départements, dont le taux d'équipement au regard de sa population est inférieur à la moyenne nationale, le suivi attentif du maillage territorial en dispositifs de recueil suivi porté par le ministe de l'Intérieur, traduit l'engagement du gouvernement à garantir un service de proximité de qualité pour tous les usagers sur l'ensemble du territoire national et à maintenir sa vigilance sur ce point, et c'est pourquoi je peux vous annoncer qu'un certain nombre d'annonces seront faites prochainement pour poursuivre cet effort national auquel nous sommes attachés pour accélérer ces procédures qui devrait ne pas dépasser 3 semaines un mois pour tout usager. Merci de votre Madame parfait, merci beaucoup, la parole est donc maintenant à monsieur Alain Milon pour sa question orale. Monsieur le Ministre, je voudrais attirer votre attention sur la modification des critères de certification environnementale des exploitations agricoles dans des pratiques particulièrement respectueuse de l'environnement, après 10 ans d'existence, et afin de respecter les exigences environnementales conditionnant les aides de la PAC, chacun s'accorde à reconnaître la nécessité d'une révision du dispositif, l'objectif est d'améliorer évidemment à la crédibilité du référentiel sur le plan environnemental et de maintenir l'attractivité de la certification on l'évolution du référentiel proposé ne répond pas aux attentes, bien au contraire, la filière viticole d'appellation d'origine contrôlée est fortement engagé dans la transition environnementale, la viticulture AOC représentent aujourd'hui la majorité des exploitations certifiées en HVE haute valeur environnementale de ce fait, l'évolution de la certification HVE représente pour elle un enjeu majeur, madame la présidente, or, si la révision proposée était retenu en l'état, elle entraînerait mécaniquement une perte de certification pour un pourcentage important de viticulteurs et donnerait un coup d'arrêt à son développement, la mise en place d'un moratoire permettrait, Monsieur le ministre d'intégrer certaines propositions d'affiliés à viticoles AOC et permettrait d'atteinte des objectifs poursuivis sans pénaliser les exploitants alors que la mise en application des nouveaux principes de fonctionnement de la HVE s'applique déjà pour partie, je vous demande, monsieur le ministre comment vous envisagez de procéder afin que le nouveau référencement ne s'avère pas contre-productif en pénalisé en pénalisant pardon nombre d'exploitations engagées dans cette démarche ou qui souhaitent s'y engager. Merci infiniment cher collègue pour votre question sur la viticulture filière qui m'est cher, vous le savez, Monsieur le Ministre, nous attendons votre réponse avec impatience monsieur Marc Fesneau Ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Milon, vous m'interrogez sur la question de la je veux d'abord dire que ça a connu un succès notamment en viticulture, il y a plus de 25000 exploitations tout en France, mais il y a beaucoup de viticulteurs qui sont engagées, vous l'avez rappelé vous-même, il y avait besoin de faire évoluer le référentiel pour le rendre plus plus fort, y compris dans les discussions que nous avions avec la PAC et c'est d'ailleurs ce qui avait partagé avec nous un certain nombre de professionnels et l'essentiel des professionnels en supprimant la voix qui était la voie dite accès économique pour se concentrer, évidemment, sur les aspects environnementaux ou ne me faites part de vos inquiétudes sur les conséquences du référentiel telle qu'il a été posé sur la table à à l'issue d'un certain nombre de réunions de concertation concernant la certification elles-mêmes repose sur un ensemble de résultats ou de moyens mis en oeuvre à l'échelle de l'exploitation permettant le déploiement de pratiques, durables, avec des objectifs environnementaux, le niveau de la nouvelle conditionnalité est tu ne donnée d'entrée du processus, il n'est pas la cible en soit par ailleurs vous m'interrogez sur la question au fond du calendrier première éléments certains avaient porté la nécessité de porter un un moratoire puisque le le dispositif devait se mettre en oeuvre dès le premier octobre 2023 nous avons accepté l'idée dans une négociation avec Bruxelles que ce que que calendrier puisse être reportée

ils peuvent aller jusqu'au bout de leur procès, c'est-à-dire au bout des 3 ans, ils pourront aller à ce moment-là, jusqu'à 2024 et donc on a bien incertain, hein, un dispositif qui a permis de consolider ce qui sont rentrés et puis un dispositif pour les nouveaux entrants, en revanche, et on l'a dit lors d'une réunion auquel vous participiez dans le Vaucluse, il y a quelques jours seulement, j'ai dit que j'étais prêt à discuter avec la filière viticole à partir du référentiel telle qu'il était posé pour regarder les impasses qui pourraient être créés, donc pas d'inquiétude pour ceux qui sont déjà dans le dispositif ah ils pourront prolonger dans la période de 3 ans, éventuellement jusqu'en 2024 et puis 2ème élément se mettre au travail pour faire en sorte qu'on trouve des solutions pratiques au sujets techniques parfois très techniques qui sont, qui sont posés, qui peuvent être un frein à l'entrée, or nous avons besoin de développer le Merci, cher collègue, vous savez, une poignée de secondes pour répliquer. Merci madame vous merci monsieur le ministre, nous acceptons évidemment volontiers votre invitation à travailler ensemble. Merci, cher collègue, la parole est à présent au sénateur Didier Rambaud pour sa question orale. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, je souhaite donc vous alerter sur la situation des producteurs de lait bio, ces agriculteurs connaissent une dégradation de leur situation depuis plusieurs mois principalement à cause d'une baisse de la consommation des produits bio, mais également d'un déséquilibre des marchés, en effet, il se trouve qu'actuellement le prix du lait est un faible niveau, parfois même en dessous du prix conventionnel, ce qui ce qui m'est évidemment les exploitations en situation de difficultés économiques a été et continue d'être aggravée par les conséquences de la sécheresse sécheresse historique de l'été 2022 le manque important du fourrage qui en résultent, pourrait engendrer de graves répercussions dans les mois à venir, à savoir des ventes partielle du cheptel ou encore des baisses de production sur mon département l'Isère que vous connaissez bien puisque vous êtes souvent venu ces derniers mois et plus particulièrement sur les zones de production des fameux fromages que sont les Saint Marcellin et Saint-Félicien, les producteurs ont jusqu'à présent réussi à maintenir le prix du lait bio en refusant des baisses de celui-ci, cependant, les producteurs font aujourd'hui face à une situation inconfortable à double titre : d'abord parce qu'ils observent que les laiteries refuse d'augmenter le prix du litre au motif de la prise de l'de l'augmentation de la prise en compte de l'augmentation des charges et dans le même temps, parce que les distributeurs constate avec stupeur que la grande distribution ou les fromageries pratique de leur côté des hausses de prix face à ce constat, l'agriculture biologique et plus particulièrement l'élevage laitier réclame des mesures pour soutenir la filière avec par exemple la permission pour les éleveurs de sortir du bio sans pénalité, le report des annuités d'emprunt, une possibilité de fixation du prix du lait ou au niveau de de de base du lait au niveau national par l'interprofession ou encore un soutien à l'achat de fourrage ou un accompagnement des exploitations les plus fragiles, notamment pour les jeunes agriculteurs, monsieur le Ministre, entre les pistes que je viens de de citer ou parmi toutes les autres, quelle mesure vous semble-t-il pertinent de prendre afin de soutenir la filière du lait bio, je vous remercie. Merci, cher collègue, Monsieur le Ministre, Marc. Nous, pour vous répondre, merci madame la présidence mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, Rambo, merci de votre question qui permet de pointer le du doigt un sujet particulier qui est le sujet du de la filière Terres bio qui souffrent assez durablement désormais d'une crise, notamment au travers du lait et de mettre en valeur aussi des zones de production comme celle que vous connaissez bien, je pense au Saint Marcelin ou au sein, Félicien, vous avez évoqué un certain nombre de mesures, la première mesure pour moi, c'est dans le cadre des négociations commerciales tous les jeudis, je tiens une réunion des négociations commerciales qui paraît parfois une réunion assez fastidieuse mais qui permet à chaque fois de mettre chacun devant ses responsabilités, en l'occurrence, ne sont pas les producteurs, qui devrait être mis devant leurs responsabilités, mais c'est les transformateurs ou la grande distribution, on a un sujet quand même de répercussion des hausses de charges pour les producteurs qui ne se refait pas chez les transformateurs ou qu'on ne retrouve pas dans la grande distribution, l'intervention d'un certain nombre de distributeurs qui ont, qui se sont dits prêts à s'engager pour une revalorisation du prix du lait, certains l'ont déjà fait, il faut désormais que dans la transformation, on puisse ensuite ça puisse se faire, et puis il y a un sujet particulier du bio qui est qui est est au au sujet de pouvoir d'achat des Français qu'on connaît bien et qui est bien documenté, qui est une baisse de la nature des produits qui sont âgés et ça touche les fromages d'origine bio et le lait bio de d'une manière plus générale première éléments essayer d'accompagner les éleveurs qui sont touchés par les phénomènes de sécheresse et c'est tous les dispositifs que j'ai annoncé d'accélération du dispositif de calamité sécheresse de pour ceux qui sont en transformation, d'avoir des dispositifs d'aide qui allège la charge pour les plus énervés intensif, on a un dispositif qui a été Renault TIFIA à Bruxelles, pour faire en sorte qu'on tienne mieux compte des réalités agricoles, y compris du cycle de production pour pouvoir mieux les accompagner et puis 3 nous permettrait, dire qu'on ne fera pas l'économie d'une réflexion globale sur la question du bio on a une croissance très forte, une croissance à 2 chiffres pendant des années et des années, on est désormais manifestement sur une décroissance voir en tout cas sur un palier, on a besoin de travailler avec l'ensemble de la filière pour faire en sorte que nous trouvions des voies et moyens de d'avancer sur ces éléments, d'abord pour mieux identifier ce qui est le bio dans le l'ensemble des références pour montrer la mise en valeur qui là et pour accompagner les producteurs et les éleveurs de faire pour faire en sorte que vous ce qui est le risque principal, qui n'est pas de décapitalisation. Merci, monsieur le Ministre, la parole est à présent à notre collègue le sénateur Monsieur Antoine Lefèvre. Merci madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, Monsieur le Ministre, les producteurs de pommes de terre ne cachent pas leur préoccupation concernant les récoltes 2022, en effet, l'été exceptionnellement chaud et sec que nous avons connu dans finit pas de révéler ses conséquences désastreuses désastreux sur notre agriculture après les viticulteurs et les producteurs de lait que nous venons d'évoquer, c'est donc désormais au tour des producteurs de pommes de terre, de tirer la sonnette d'alarme sur les pertes prévisionnelles sur la prochaine campagne de récolte leur filière accusera cette année une baisse de moyenne de 20 de son rendement en raison des effets de chaleur sur les cultures, avec des chiffres encore plus dramatique pour les producteurs qui ne disposent pas de système d'irrigation, en août, en ajoutant à cela des effets sur l'inflation de l'inflation sur les coûts de production et l'exploitation des tarifs de l'énergie, c'est une baisse sans précédent de la superficie totale cultivée qui devrait poindre en 2023, l'Union nationale des producteurs de pommes de terre que vous aviez au ministère de l'Agriculture au début du mois de septembre, a exprimé le souhait d'un dispositif de sauvegarde soit mises en oeuvre, qu'il soit placé sous la forme d'un prêt garanti par l'État, engagé sur les seules surfaces plantées en 2023 et remboursable en fin de campagne, une hausse des ZZ couplé à hauteur de 500 euros par hectare serait ailleurs par ailleurs susceptible de sauver de la faillite, nombres de petits producteurs pris à la gorge par l'accumulation des imprévus, le régime universel d'indemnisation sur les pertes de récoltes résultant d'aléas climatiques prévues par la loi du 2 mars 2022, sur laquelle le Sénat a très largement marqué son empreinte aurait amplement suffi à compenser les pertes et assurer une protection salutaire aux agriculteurs, celui-ci ne prendra pourtant effet qu'à compter du 1er janvier 2023, soit à peine plus de 4 mois trop tard pour couvrir les pertes subies à l'été 2022 par les producteurs assuré quels instruments transitoire pourrait donc mis en place pour compenser les pertes des producteurs de pommes de terre, je vous remercie. Merci, cher collègue, j'invite monsieur Marc Fesneau Ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire à vous répondre. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Lefèvre merci de cette question qui vient éclairer d'un nouveau jour, vous l'avez dit 3ème filière 3ème filière où on évoque au fond les difficultés liées aux aléas climatiques, de dérèglement climatique, j'ai rencontré effectivement le les organisations de producteurs de pommes de terre, moi personnellement, et mon cabinet pour faire en sorte d'être et de d'essayer de trouver une voie et un chemin d'abord dire quand même que sur la production, les nouvelles sont moins mauvaises que nous que l'on ne au démarrage, l'inquiétude, vous l'avez dit, c'est l'inquiétude pour l'année prochaine, c'est la remise en culture, qui pourrait être une vraie difficulté puisque la production va diminuer quand même nos évaluations font état de moins 9 % par rapport à 2021 et moins 6,5 pour 100 par rapport à la moyenne quinquennale et donc, si ça ne nécessite plusieurs éléments de réponse donc sur la sécheresse, compte tenu du du règlement de la récolte, un nouvel examen de la situation va être privilégiée dans les prochaines semaines pour regarder ce qui peut être indemnisés par les dispositifs classique pour le 2ème sujet vous avez évoqué le PG, on en a, on y a travaillé avec les services de Bruno Lemaire Éric Bruno Lemaire, on ne trouve pas la voix pour être très clair avec vous sur le PGE parce que là on ouvrirait une boîte le PGE a été bien identifiée pour Covid et pour résilience Ukraine mais là on est sur un sujet climatique qui ne paraît pas rentrer et, par ailleurs, nous serions amenés à rentrer d'autres filières, ce qui serait une difficulté supplémentaire, je veux dire simplement qu'on les a orientés et j'ai demandé qu'on puisse expertiser le fait qu'il puisse rentrer en revanche vers Le Pecq résilience qui est doté d'une enveloppe de 150 millions d'euros et qui leur permettrait de faire face à cette à ces éléments, je continue à travailler aussi à des solutions par rapport aux augmentation des coûts énergétiques, il vient de produire un effet ciseau et je le disais tout à l'heure, on est en cours de notification d'un régime d'aide qui permettra notamment sur les sujets de réfrigération le maintient au frais des de de ses récoltes pour les producteurs de pommes de terre, enfin, je voudrais dire un dernier mot, parce que je pense que ça c'est un élément ça c'est les éléments de court terme, puis sur moyen long terme, vous avez parlé de l'assurance-récolte je voudrais saluer le travail qui a été fait, effectivement, en particulier au sénat pour mettre en place un dispositif qui robuste dans un temps assez record puisque loi au mois de mars, mise en application au 1er janvier mais ça ne concerne pas ceux qui sont touchés cette année, en revanche, il faut qu'on travaille aussi sur un autre sujet me semble-t-il, c'est la question de la l'accès à l'eau parce que c'est la meilleure résilience est aussi l'accès à l'eau pour éviter ce que simplement l'assurance viennent se substitue substituer à des difficultés, comme celle que nous rencontrons cette année. Merci, monsieur le Ministre, chers collègues, vous avez une poignée de secondes pour réplique. et encore un petit effort à faire sur ce sujet pour qu'on puisse vraiment voir l'avenir et et notamment la l'exercice 2023 2 sous de bons auspices merci. Merci enfin la parole est donnée un autre collègue sénatrice Madame Else Joseph. Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, je m'interroge sur les conséquences de l'application de certaines dispositions prévues par la loi du 30 octobre 2018 dites Egalim en effet, au regard des témoignages locaux, elles peuvent poser de sérieux problèmes dans le domaine de la restauration scolaire et collective, tout d'abord, l'obligation d'un menu végétarien, ainsi que celle d'un approvisionnement fixé à 50 pour 100 en Reyhanli montèrent dites durable constituent de véritables difficultés, elle se heurte aux habitudes socio-culturels, des habitants qui, par exemple, continuer à donner une importance à la consommation de viande et ne sont pas toujours familiers de l'alimentation bio, l'application d'un repas végétarien hebdomadaire est une solution trop rigide et devrait davantage relever de l'incitation, il a de de la démarche volontaire que de l'obligation, on a également constaté une augmentation des déchets avec la mise en place des menus végétariens, ce qui a malheureusement entraîner une relance du gaspillage alimentaire les filières bio ne sont pas toujours suffisantes dans certaines parties du territoire français, c'est le cas dans mon département des Ardennes en raison de cette offre limitée l'approvisionnement va se faire auprès de grossistes qui recourt en même, en général, donc à des produits importés, cette situation est paradoxale, alors que l'on affirme en même temps vouloir relocaliser les approvisionnements, comme on peut le constater, les produits bio, durable, coûte plus cher et peuvent fragiliser les syndicats intercommunaux intercommunaux à vocation unique vocation multiple et Sivu Sivom qui risque de devoir augmenter les tarifs au détriment des familles et aussi des finances des collectivités locales, monsieur le Ministre, qu'envisagez-vous pour que des adaptations locales soit trouvée pour des dispositions pour les dispositions de la loi Egalim qui constituent de véritables problèmes financiers pour nos collectivités. Si cher collègue, la parole est à monsieur Marc Fesneau Ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice d'abord merci de me poser cette question qui permet de refaire un point général sur ces questions alimentaires qui sont des questions importantes, j'ai moi-même été maire et président de communauté de communes, donc je vois les difficultés à laquelle vous pouvez faire référence l'objectif et comme vous le savez, d'améliorer, avec un taux le la qualité des repas avec un taux d'approvisionnement de 50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % vous l'avez rappelé de produits biologiques, vous évoquez les difficultés que peuvent susciter les menus végétariens, il me semble d'abord que les recettes végétariennes sont assez nombreuses pour qu'on puisse avoir une panoplie qui évite le gaspillage, je pense aux aux produits laitiers pour favoriser l'introduction d'ingrédients que les jeunes enfants ont moins l'habitude de consommer mais qui consommeront néanmoins qu'ils laisseront pas sur le côté de l'assiette, vous dites quelque chose d'ailleurs qui est très juste sur le le gaspillage alimentaire mais globalement on a un sujet de gaspillage alimentaire dans la restauration scolaire sur lequel il faut que nous travaillons et parfois dans ces projets d'alimentation durable, on arrive à à travailler sur ces questions de non-gaspillage alimentaire j'ai visité un lycée agricole qui avait beaucoup travaillé sur ces questions et qui avait réussi à la fois faire évoluer vers des produits de qualité et en même temps de à lutter contre le gaspillage alimentaire 3ème élément, il y a parfois des problèmes de logistique, c'est un peu ce que vous dites, c'est le côté pratique, c'est d'arriver à trouver des producteurs dans le dans notre affaire, c'est un peu la poule et l'oeuf, si vous me permettez cette expression, on a besoin de faire en sorte que des filières comme celles-là se développent et par parfois les filières tarde, pour des tas de raisons, y compris de logistique bien légitime à se mettre en oeuvre, il me semble que dans ce cadre-là, d'ailleurs les plans alimentaires territoriaux peuvent être un outil pour mieux coordonner la demande pour faire en sorte que vis-à-vis des Sivu des Sivom, des communes ou des intercommunalités qui exerce la compétence, il puisse trouver une offre qui permettent de répondre à un cahier des charges qui permet aussi aux agriculteurs de répondre parce qu'on sait comment la logistique peut se développer, je voudrais saluer quand même, il y a beaucoup d'initiatives qui se prennent dans les collectivités, qui font en sorte d'essayer d'aller sur ce chemin, dernier point, il me semble que je voulais vous dire qu'on a mis en place, y compris dans le plan de relance des des mécanismes de soutien aux collectivités pour faire en sorte qu'elle puisse mettre à niveau leur cantine parce que la restauration de proximité, c'est aussi une question d'investissement pour les collectivités donc on va regarder comment on peut poursuivre ce travail là, dans les années qui viennent pour essayer de mettre en meilleure adéquation l'offre et la demande. Merci, Monsieur le Ministre, vous avez une poignée de secondes, si vous souhaitez répliqué chers collègues. les collectivités. Merci, monsieur le Ministre, mes chers collègues, je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 14 heures 30 pour l'examen du projet de loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, la séance est suspendue, bon appétit.

Merci,